d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site

et indépendants. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le mécontentement du monde agricole vient de loin.

vous avez répondu à ce mécontentement, monsieur le Premier ministre, en vous rendant notamment en Occitanie et dans d’autres territoires pour apporter des réponses. Certaines solutions ont été mises en œuvre immédiatement : je pense au

l’agriculture pour échanger avec les agriculteurs, leurs représentants, les éleveurs, les pêcheurs, comme je le fais constamment depuis ma nomination en tant que Premier ministre au début du mois de janvier.

J’ai échangé avec les représentants des syndicats agricoles. Il y a trois semaines, les principales organisations ont annoncé qu’elles levaient leurs barrages à la suite des engagements très concrets que j’ai pu prendre au nom du Gouvernement, en lien avec mes ministres, Marc Fesneau, Agnès Pannier Runacher, Christophe Béchu et Bruno Le Maire.

Les extrémistes, travestis en colombes, auraient sans aucun doute appelé à l’envoi de troupes pour soutenir la Russie s’ils étaient aujourd’hui au pouvoir. Non seulement l’argent du mage du Kremlin les a financés, mais l’alliance avec la Russie figurait en toutes lettres dans leur programme. La France n’est pas en guerre au sens où nous l’entendions au XX siècle, mais elle sait très bien qu’une large part de sa propre sécurité et de celle du continent se joue à l’Est. Laisser gagner Poutine, c’est accepter la défaite de nos valeurs. Notre groupe ne peut s’y résoudre et se félicite que le Parlement soit amené très prochainement à voter sur le sujet.

ce type d’actions de guerre 4.0, nos adversaires cherchent à saper notre volonté, voire à nous imposer la leur. Dans ces conditions, il nous faut déployer davantage de moyens pour prévenir et contrer ces influences et ces cyberattaques, tout en préservant la liberté de nos concitoyens. Nous ne réussirons pas sans eux. Lucidité, formation et participation des citoyens sont primordiales pour la robustesse de notre démocratie. Beaucoup reste à faire dans ce domaine. La France doit continuer à soutenir l’Ukraine dans son combat pour rester souveraine. C’est un impératif. Nous devons bien sûr assurer les livraisons d’armes, mais il nous faut aussi renforcer notre arsenal. Monsieur le ministre, dans le champ informationnel,

ukrainien, qui résiste avec une bravoure qui fait l’admiration du monde entier. Depuis quelques mois, la posture du régime s’est durcie à la fois sur la ligne de front, ligne de front, le territoire ukrainien, en Russie – avec l’assassinat politique d’Alexeï Navalny, qui aura donné sa vie pour la liberté, et dont nous saluons la mémoire mémoire –, en Europe et en France, qui sont désormais la cible de vastes campagnes de manipulation et de désinformation orchestrées par des intérêts ou des courroies de transmission russophiles, qui veulent porter atteinte à notre débat public. L’intention de Vladimir Poutine est double

Le 12 janvier dernier, Stéphane Séjourné, avec ses homologues allemand et polonais, a révélé l’existence de 193 sites dormants destinés à perturber le débat public et les futures élections, grâce au travail remarquable de Viginum, le par la volonté du Président de la République, et placé sous l’autorité du Premier ministre. Ce lundi 26 février, à Paris, Emmanuel Macron a convoqué un sommet international, qui a rassemblé vingt sept chefs d’État et de gouvernement ou leurs représentants directs. Les manœuvres informationnelles étaient à l’agenda de cette conférence et feront l’objet d’une réunion de suivi par les ministres des armées et des affaires étrangères. Pour ma part, j’ai appelé la Commission européenne à se saisir des pouvoirs qui sont les siens aux termes du règlement sur les services numériques pour obtenir de la part des grandes plateformes un engagement ferme,… Il faut conclure ! … celui de faire respecter le silence électoral lors des élections européennes des 6 et 9 juin prochains.

Le groupe auquel j’appartiens, le RDSE, n’a pas la réputation de compter dans ses rangs des extrémistes ou des excités. Ça non ! Il s’agit du plus ancien groupe politique du Sénat, qui s’appuie sur les valeurs essentielles, au rang desquelles on trouve la défense des principes républicains, fondements de notre démocratie. Groupe minoritaire dans cette assemblée, il ne s’oppose jamais par principe au Gouvernement ni à la majorité sénatoriale. À la tribune, lors des explications de vote sur le projet de loi de finances pour 2024,

main. Avec la publication du décret du 22 février 2024 portant annulation de près de 10 milliards d’euros de crédits votés en loi de finances, vous brutalisez la démocratie ! Dans notre République, il revient en effet au Parlement de voter le budget.

en affichant le même mépris et la même assurance, vous avouez en réalité avec ce décret que vos prévisions budgétaires étaient fondées sur des hypothèses trop optimistes, et cela malgré nos multiples mises en garde.

ce n’est pas la France qui le dit : au même moment où nous revoyons nos prévisions de croissance, la Commission européenne,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, redonner aux prix leur rôle de signaux de marché, tel était le mot d’ordre des réformes de la politique agricole commune de 1992 et 1999. plus tard, nous y sommes : les prix garantis ont disparu ; les prix sont volatils et singulièrement bas dans plusieurs secteurs de production agricole. Initialement, les aides directes sont attribuées pour compenser ces baisses de prix. Au fil des réformes, elles sont de plus en plus découplées des facteurs de production, mais restent majoritairement liées à la surface des exploitations. Madame la ministre déléguée, il y a quelques semaines, le Gouvernement exprimait son refus de mettre en œuvre l’une des principales revendications du monde agricole, celle d’une meilleure régulation des prix. Acculé par les mobilisations des agricultrices et des agriculteurs, le Président de la République a fini par reconsidérer la question et propose désormais un prix plancher. Madame la ministre, il va de soi qu’un prix plancher national renforcerait mécaniquement les importations en provenance du reste de l’Europe et des pays tiers. Vous le savez, pour être efficace dans notre marché unique, ce prix garanti doit être européen. Alors, comment comptez vous négocier cette unification des prix garantis à l’échelle européenne ? Sur quels critères, pour quelles productions, et selon quel calendrier ?

envisageons d’aller un cran plus loin, c’est à dire de construire les prix sur les indicateurs de référence – c’est l’esprit de la loi Égalim – qui sont élaborés par les filières, en faisant en sorte que cette construction « marche

pour discuter de ces sujets, notamment des enjeux de régulation. chers collègues, ma question s’adressait à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Les passions populaires que suscite chaque année le salon de l’agriculture ne doivent pas nous faire perdre de vue la crise structurelle que traverse

les grands actionnaires des industries agroalimentaires captent la moitié de la valeur ajoutée, après paiement des salaires et des impôts de production.

Aujourd’hui, certains grands groupes industriels du secteur se livrent à un véritable chantage, allant jusqu’à menacer de refuser de collecter le lait auprès des producteurs qui n’accepteraient pas le prix qu’ils imposent. Dans un tel contexte, comment ne pas comprendre que l’accumulation des normes et des paperasseries ajoute à l’exaspération, même si ce ne sont pas elles qui contribuent à diminuer le revenu paysan

Vous relayez ici la colère légitime de nos agriculteurs, et vous avez raison ! Il nous faut répondre à cette colère et apporter des solutions concrètes à ces femmes et à ces hommes qui consacrent leur vie à nous nourrir, une vie d’efforts et de contraintes, qui doit être justement rémunérée.

heures lundi soir quand, à la sortie de la conférence internationale de soutien à l’Ukraine, le chef de l’État a déclaré que l’envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne devait pas être exclu. Les Français découvrent alors, en direct, un changement fondamental de notre stratégie, au travers du soutien que nous apportons à l’Ukraine face à l’invasion d’une partie de son territoire par la Russie. Cette déclaration est d’autant plus incompréhensible qu’elle remet en cause toute la cohérence défendue jusqu’ici par la France. Mais que signifie cette initiative dont nos propres alliés au sein de l’Otan se sont aussitôt désolidarisés ?

Alors, monsieur le Premier ministre, quels engagements votre gouvernement prend il ici pour respecter l’ordre constitutionnel et continuer de défendre notre intérêt le plus fondamental, à savoir la paix ?

pour la sécurité de l’Union européenne et de la France. En effet, chacun sait que les dictateurs ne prennent pas de vacances et que, si l’Ukraine devait tomber – mais nous ferons tout pour l’éviter –, la ligne de front se déplacerait inévitablement vers l’ouest. Quand la maison du voisin brûle et que l’incendie menace de se propager, on ne reste pas les bras ballants ; on se lève et on agit ! Comme le disait Raymond Aron en 1939, nous croyons à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c’est qu’elles le veuillent. C’est la raison pour laquelle le Président de la République a convoqué, lundi 26 février, un sommet international auquel vingt sept chefs d’État et de gouvernement, ou leurs représentants directs, se sont rendus ils se sont entendus pour poursuivre notre soutien à l’Ukraine, pour faire plus, mieux et différemment. À cette occasion, le Président de la République a déclaré que nous ne pouvions rien exclure, que nous devions explorer tout le champ des possibles, tout en accroissant notre soutien à l’Ukraine. Ce serait une faute grave et une menace pour notre sécurité que de refuser de débattre de toutes les options qui se présentent à nous, aujourd’hui

chargé des comptes publics, vous avez décidé par décret d’une nouvelle cure d’austérité de 10 milliards d’euros pour notre pays, reconnaissant par là même le caractère insincère du projet de loi de finances pour 2024. Depuis sept ans, vous voulez faire croire aux Français que l’on peut réduire, à la fois, les recettes fiscales de l’État et les dépenses publiques. Or, dans le domaine des finances publiques, moins plus moins ne fera jamais plus Alors qu’un gouvernement devrait protéger et anticiper l’avenir, vous participez aveuglément au creusement des inégalités dans notre pays et vous précarisez, encore et toujours, les plus fragiles.

en 2024. Emploi et formation : – 1,1 milliard d’euros, et autant de demandeurs et demandeuses d’emploi sans solution de formation et de retour vers l’emploi. Pourtant, l’argent est là. Il existe. Niches fiscales et sociales, réductions d’impôts, baisses des cotisations patronales, aides directes : pour les grandes entreprises, pour les actionnaires, pour les 1 % les plus riches de notre pays, l’argent pleut chaque année un peu plus, mais mais sans aucun effet manifeste sur les indicateurs économiques qui vous sont si chers. Monsieur le ministre, quand allez vous abandonner ce dogme absurde et inefficace du « toujours moins de fiscalité pour les plus aisés », au détriment des services publics et des réponses urgentes et pérennes à la crise sociale et climatique ? Quand allez vous cesser de mentir aux Français en prétextant une conjoncture défavorable que vous étiez le seul à ne pas voir venir ? Quand allez vous enfin anticiper et investir pour l’avenir ?

Monsieur le Premier ministre, le chef de l’État a tenu lundi dernier des propos qui ont surpris, voire inquiété, les Français et nos alliés. En juin 2022, il recommandait de ne pas humilier la Russie, alors que les Ukrainiens subissaient depuis cent jours les assauts de l’armée russe. Aujourd’hui, il affirme que l’envoi de troupes au sol ne devrait pas être exclu. Il a compris que la méthode douce ne fonctionnait pas avec Vladimir Poutine. Son entourage tente d’expliquer, d’ailleurs, qu’il aurait souhaité envoyer un signal à la Russie. Mais on ne peut pas improviser sur un tel sujet sans se concerter avec nos alliés Ces effets de manche nous isolent et ils obligent nos alliés à se désolidariser. Le sujet est trop sérieux et trop grave : c’est de la sécurité des Français et de l’Europe qu’il s’agit. Monsieur le Premier ministre, comment le chef de l’État peut il sérieusement envisager l’envoi de militaires sur le terrain alors que nous ne sommes qu’au début de la relance de notre effort de défense ? Comment imaginer envoyer des troupes au sol, alors que nous ne sommes pas capables de fournir à l’Ukraine les armes et les munitions dont elle a besoin ? Je terminerai mon propos par ces mots du Premier ministre polonais, Donald Tusk : « Si tous les pays de l’Union européenne étaient autant impliqués dans l’aide à l’Ukraine que la Pologne, il ne serait sans doute pas nécessaire de discuter d’autres formes de soutien. » La

D’abord parce que, derrière l’Ukraine, il y a nous ! Si un certain nombre de pays historiquement neutres – je pense à la Suède, à la Finlande – font le choix de rejoindre l’Otan, c’est bien parce qu’ils perçoivent une menace directe à leur

l’emporte : la guerre que mène ce pays contre l’Ukraine est aussi une guerre contre un modèle et des valeurs qui sont les nôtres. La Russie cherche à démontrer que la démocratie serait un état de faiblesse et que l’État de droit serait un état d’indécision.

Monsieur le Premier ministre, le 19 février dernier, vous avez choisi d’envoyer le ministre de l’économie et des finances, M. Bruno Le Maire, sur un plateau de télévision pour annoncer

Le ralentissement économique a probablement démarré à la fin de l’année 2023, avec un impact sur les recettes en 2023 et donc probablement – nous le saurons à la fin du mois de mars – un impact sur le solde public de l’année 2023.

nous n’aurions pas de problème pour équilibrer nos politiques publiques. Donc oui, il faut continuer à inciter au travail et assumer la recherche d’un modèle social moins coûteux et plus efficace ; cela fait partie de nos pistes de travail. Je sais, monsieur le rapporteur général, que vous y travaillerez avec nous lors des prochains mois. La parole est à M. Jean François Husson,

Oui, vous avez choisi de doper la croissance dans vos prévisions macroéconomiques, à hauteur de deux fois ce qu’avait prévu le consensus des économistes. Vous êtes donc, finalement, rattrapé par la patrouille et par une forme de mise en danger ou d’amateurisme.

après des semaines de tension dans le monde agricole et des années de frustration à la suite des échecs successifs des lois Égalim, le Président de la République semble, à la surprise générale, avoir enfin entendu la principale revendication portée par les paysans : la juste rémunération de leur travail. Pourtant, comme nous le constatons avec le flou gouvernemental qui perdure depuis samedi, cette mesure du prix plancher, qui pourrait être une bonne idée, risque de malheureusement rester au stade de la grande promesse. La véritable question que nous devons nous poser est la suivante : comment remettre du revenu dans nos fermes, et tout particulièrement dans les filières et les régions les plus impactées Le plan de trésorerie d’urgence, avec de simples demandes de moratoire aux banques, ne supprimera pas cette pression financière. L’annonce d’une nouvelle loi Égalim – la cinquième du nom ! –, dont une entrée en vigueur ne saurait être envisagée avant la fin de 2024, semble une réponse bien incertaine et lointaine face à l’urgence actuelle. Comme avait pu le faire Jean Glavany, avec les contrats territoriaux d’exploitation (CTE), qui ont sauvé de nombreuses fermes, il est nécessaire de penser à un dispositif plus adapté aux enjeux d’aujourd’hui et aux réalités des territoires. Les inégalités entre les filières et les régions, voire entre deux exploitations situées à quelques kilomètres, poussent à une contractualisation territorialisée et individualisée. Pour permettre cela, madame la ministre, le groupe la ministre, le groupe socialiste du Sénat vous demande d’engager solennellement une révision du plan stratégique national (PSN) de la politique agricole commune (PAC). Ces révisions nationales sont rendues possibles par la dernière PAC, et peuvent nous donner des moyens d’agir : une meilleure régulation du prix ; une plus juste répartition des aides publiques, notamment en renforçant les paiements distributifs aux premiers hectares et en accompagnant davantage la transition agroécologique ; et enfin, un soutien aux filières en difficulté, qui façonnent et font vivre nos territoires.

traverse une crise majeure, sans doute l’une des plus importantes de ces dernières décennies. Le covid 19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, associée à la déstabilisation des marchés énergétiques et agricoles organisée par M. Poutine, ou encore le dérèglement climatique et les menaces qu’il fait peser sur nos récoltes et la biodiversité, sont autant de sources dans lesquelles cette crise trouve ses racines. Dans ce contexte, il est naturel que la colère de nos agriculteurs s’exprime haut et fort. Pour reprendre les mots de Georges Clemenceau, la colère gronde, mais elle ne doit pas rester sourde aux appels de l’action. Comment pourrions nous tolérer que ceux qui nourrissent notre nation ne puissent vivre décemment de leur labeur ? C’est pourquoi le Gouvernement est à l’action pour traiter le problème fondamental de la juste rémunération, pour les protéger de la concurrence déloyale venant de pays qui n’appliquent pas les mêmes règles environnementales que les nôtres, les nôtres, pour simplifier leur vie, afin qu’ils puissent passer plus de temps sur leur exploitation et moins dans leur bureau – c’est aussi une façon d’alléger leurs charges. Avec Marc Fesneau, je suis en permanence sur le terrain, au contact et à l’écoute des agriculteurs. Nous n’avons pas attendu le salon de l’agriculture pour agir. C’est ainsi que, sous l’égide du Président de la République et du Premier ministre, nous déployons déployons rapidement un plan d’action pour répondre point par point à leurs difficultés. Les fonds d’urgence ont d’ores et déjà été mis en place et les premiers paiements ont été effectués depuis mi février, comme nous nous y étions engagés.

Nous avons également négocié hier, avec le ministre de l’économie, des mesures de trésorerie avec les banques. Et le PSN ! Les premiers textes de simplification ont été établis. Certains sont d’ores et déjà publiés. Nous engageons dès à présent une réflexion, la mission Égalim qui va être confiée aux députés Alexis

! Nous n’avons pas de raison de le réviser à ce stade, puisque nous avons un plan d’action adapté à la situation.

le Président de la République, survolté, en bras de chemise, dans un grand numéro de communication comme il les affectionne tant, annonçait… – tadam Sortie de nulle part, réclamée par personne – nous l’avons vérifié avec la présidente Estrosi Sassone au salon de l’agriculture –, cette annonce a laissé sans voix les paysans et les organisations professionnelles. Vous même aviez du mal à cacher votre stupéfaction.

Oui, les prix planchers relèvent de l’économie administrée et n’ont aucun sens dans un marché ouvert. Mis en œuvre, ces prix deviendront des prix plafonds.

un soutien structurel, même aux filières les plus fragiles comme celle de l’élevage. Surtout, cette méthode jupitérienne casse toujours et encore cette confiance qu’il faut recréer entre la parole publique et le monde agricole. Ma question est donc simple : que diable êtes vous allée faire dans cette galère des prix planchers,

des réformes permettant de mieux rémunérer nos agriculteurs. Il s’agit des lois Égalim, dont j’ai longuement parlé dans mes dernières réponses. Nous avons fait évoluer le rapport de force dans la négociation entre agriculteurs, industriels et distributeurs, mais le compte

le prévoyaient les lois Égalim : en faisant en sorte que le prix soit négocié sur la base d’indicateurs de référence entre agriculteurs et industriels avant que la négociation ne démarre entre industriels et distributeurs.

l’effondrement de nos exportations, et un risque d’augmentation des importations.

le dérèglement climatique va profondément bouleverser – cela commence déjà – nos modes de vie, particulièrement dans les territoires de montagne. Comment accompagner la transformation dans ces territoires ? J’ai lu récemment deux rapports.

Les magistrats de la rue Cambon dépeignent un secteur d’activité sous perfusion de fonds publics, « incapable » de s’adapter aux enjeux écologiques. Leur conclusion générale se fonde exclusivement sur une grille de lecture financière et sur des indicateurs très contestables. À titre d’exemple, la Cour des comptes évalue la vulnérabilité des stations sur la base d’une altitude moyenne sans prendre en compte l’étendue du domaine, l’exposition des pistes ou encore le nombre de communes supports. À croire que la culture montagnarde des magistrats de la Cour des comptes se limite à la montagne Sainte Geneviève et ses 61 mètres d’altitude à Paris ! Ma question est simple, madame la ministre : pour quelle vision de la montagne le Gouvernement va t il opter ?

des projets très concrets avec des subventions massives de plusieurs millions d’euros pour aménager aujourd’hui la montagne et faire en sorte que celles qui seront moins enneigées puissent proposer d’autres activités. Je tiens à rappeler que les clients

complètement à côté de la plaque si l’on regarde la manière dont les choses ont été évaluées. Il faut que cela soit dénoncé clairement par le Gouvernement. Par ailleurs, nous attendons une nouvelle version du plan d’aménagement de la montagne,

pour le groupe Les Républicains. Madame Belloubet, vous avez été récemment nommée ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse à la suite de vos prédécesseurs qui se sont succédé à un rythme soutenu, voire trop soutenu, ce qui témoigne de l’absence de politique éducative du Président de la République. Quel point commun entre Jean Michel Blanquer et Pap Ndiaye ? Nous avons vite compris que le second avait à cœur de remettre en cause l’action du premier… Vous succédez à Gabriel Attal qui avait, en son temps, fait des annonces. Allez vous à votre tour remettre en question ces engagements ? J’ai quelques interrogations êtes vous favorable, comme lui, au redoublement et à l’aménagement du collège unique, avec la mise en place de groupes de niveau et non de groupes flexibles ? Êtes vous pour la généralisation de la tenue scolaire, de l’interdiction de l’abaya et pour le respect de la laïcité lors des sorties scolaires ? Êtes vous pour la restauration de l’autorité à l’école, ou s’agit il toujours de « fariboles », pour reprendre vos anciens propos ? Enfin, madame la ministre, alors que votre prédécesseur a toujours indiqué que l’éducation nationale était la mère des batailles, comment pouvez vous justifier la baisse de près de 700 millions d’euros des crédits de l’enseignement scolaire ? Éclairez nous sur le projet que vous voulez mettre en œuvre pour enrayer la baisse de niveau des petits Français

Grosperrin, le Président de la République et le Premier ministre ont fixé ce qu’étaient nos priorités pour l’école. D’une part, clairement, améliorer nos résultats scolaires et donc l’efficacité de notre système éducatif, un objectif qui me semble me semble partagé par les uns et les autres ici. D’autre part, assurer le bien être de nos élèves et de nos enseignants dans l’école. Il me semble qu’un climat de sérénité scolaire est indispensable pour la réussite éducative. Ce n’est pas la question ! Pour le reste, vous me posez une série de questions, dont certaines m’étonnent. Vous me demandez si je suis favorable à la laïcité. Quelle autre réponse pourrais je vous apporter qu’une réponse positive ? La laïcité est indissolublement liée à la République.

orientations qui ont été fixées par mon anté prédécesseur, M. le Premier ministre, autour du choc des savoirs. Évidemment, je vais le faire, car cela constitue une série de mesures qui sont indispensables pour la réussite de nos élèves. Je veillerai, dans le cadre d’un dialogue avec les représentants des personnels, des parents, de l’ensemble de la communauté éducative, à rendre ces mesures parfaitement applicables dès la rentrée prochaine. C’est mon ambition. Enfin, un dernier mot sur le budget de l’éducation nationale, qui représente à peu près 64 milliards d’euros, pensions non comprises. Les annulations de crédits que nous devons supporter – nous le faisons parce que c’est un effort collectif nécessaire à la stabilité financière de notre pays – représentent à peine 1 % de l’ensemble des annulations budgétaires, soit 683 millions d’euros. Nous ne supprimerons aucun poste. Nous resterons fidèles aux choix que nous avons faits pour la rentrée prochaine. C’est mon ambition

l’air faussement grave, la nécessité de réaliser 10 milliards d’euros d’économies sur le budget pour 2024. Cette annonce inédite, départie de toute onction démocratique, et dont je viens de rappeler le montant colossal, a opportunément permis, une fois de plus, de se détourner du Parlement.

Votre prévision de 1,4 % était irréaliste, tout comme celle retenue de 1 %. On frôle l’insincérité budgétaire ! Monsieur le ministre, l’austérité n’est pas une fatalité : c’est un choix politique. En refusant d’augmenter les impôts des plus aisés, vous faites le choix d’une punition collective à l’égard des classes moyennes que vous prétendez pourtant servir. Alors que le quinquennat du Président de la écologique ou ne sera pas », il est stupéfiant de constater que, avec plus de 2 milliards d’euros de coupes sèches, le budget le plus impacté reste celui de l’écologie. Sans parler des 400 millions d’euros de dotation du fonds vert que vous supprimez pour nos collectivités territoriales Loin des discours vertueux qui ne convainquent plus personne, une fois de plus, c’est l’écologie qui fera office de variable d’ajustement. d’ajustement. Alors que l’effet récessif de cette suppression de crédits est établi, pensez vous qu’un tel coup de rabot budgétaire soit de nature à réarmer l’économie que vous prétendez défendre ?

Permettez moi de revenir sur les prévisions économiques. Le dépôt du projet de loi de finances a eu lieu le 27 septembre dernier. À cette époque, l’OCDE,

En novembre dernier, la Commission européenne prévoyait encore une croissance de 1,2 %. Votre accusation d’insincérité serait valable si nous étions seuls à revoir notre prévision de croissance durant ce mois de février. Or, je vous l’ai dit, la Commission européenne, l’Allemagne et nous mêmes avons tenu compte des effets du ralentissement de la conjoncture

Il faut conclure. Mais en supprimant 8 000 postes dans l’enseignement scolaire, 7 500 dans la recherche, 300 dans la justice, c’est l’avenir de notre pays que vous sacrifiez sur l’autel des marchés financiers que vous entendez contenter.

où les compensations se réduisent à peau de chagrin et surtout où les sacro saintes normes deviennent légion à la moindre esquisse de projet, il est grand temps de s’inquiéter sur la capacité à maintenir le cap. Peut on se questionner sur le rapport qualité prix de nos politiques publiques – et ce n’est plus un gros mot ? Selon l’OCDE, le coût annuel français d’un élève dans le secondaire est de plus de 13 000 dollars pour une moyenne de 11 000 dollars dans le reste des pays membres de l’organisation internationale. Un coût en constante augmentation pour une évolution inversement proportionnelle dans le classement Pisa… Par ailleurs, le Premier ministre vient d’annoncer la suppression de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour 2024 : les bénéficiaires auront donc accès au À toutes fins utiles, je vous indique que l’ASS était financée par l’État et que le RSA l’est par les conseils départementaux. Serait ce une nouvelle délégation sans moyens associés ?

solidaires de notre ferme France, laquelle gronde et s’enflamme, et cela n’a rien à voir avec l’année olympique ! Ma question est donc la suivante : allons nous vers une asphyxie programmée des départements, monsieur le ministre

Ils font face à ce qu’on appelle un effet ciseaux, que vous avez bien décrit, c’est à dire des dépenses qui augmentent et des recettes qui connaissent des difficultés. Vous avez cité les DMTO, qui baissent de 20 % environ. Certains départements en situation difficile – j’insiste sur le mot « certains » parce que la situation est très hétérogène –, et ils maintiennent leur niveau de trésorerie. Face à cela, le budget pour 2024 prévoit un certain nombre de mesures que je tiens à rappeler pour expliquer comment nous nous tenons aux côtés des départements pour ne pas les laisser seuls

d’autonomie. Le fonds national de péréquation des DMTO – un fonds de péréquation entre départements que vous connaissez – s’élève à 245 millions d’euros. Enfin, nous avons permis aux départements de s’assurer eux mêmes, avec un mécanisme qui leur permet de mettre en réserve

Union Centriste. Madame la ministre, la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR) engagée par la loi de finances pour 2024 afin de remédier aux carences de l’actuel zonage, à bout de souffle depuis sa création en 2015, est malheureusement loin de faire l’unanimité dans les territoires. De nombreux élus locaux, que je rencontre dans mon territoire et dans d’autres, parlent même déjà d’un fiasco en raison de nombreuses aberrations du nouveau régime de zonage et des inégalités territoriales qui subsistent, voire s’aggravent. Comme expliquer en effet qu’une commune de plus de 25 000 habitants soit classée, alors que de nombreuses communes rurales de très petite taille sortent du classement ? C’est la définition même de la ruralité qui me paraît ici être en jeu. Le constat est alarmant. Des départements entiers voient leurs communes sortir du classement, à l’instar de la Moselle ou du Rhône, et d’autres, partiellement, comme la Haute Loire ou le Jura. C’est peu dire que cette réforme produit du désespoir. À l’automne dernier, à plusieurs reprises, Rémy Pointereau, Louis Jean de Nicolaÿ, Didier Mandelli et moi même avions alerté quant au danger d’un classement à la maille intercommunale et aux effets pervers d’un nombre trop réduit de critères. Vous avez passé outre notre mise en garde, ce qui illustre à merveille l’adage cher au président Edgar Faure : « C’est un grand tort d’avoir raison trop tôt. » Nous n’étions pourtant pas des devins, mais simplement à l’écoute des territoires, car, jusqu’à preuve du contraire, le dialogue est plus efficace pour appréhender les difficultés territoriales que les tableaux Excel de l’administration ou la politique des algorithmes. Ma question est donc simple : que comptez vous mettre en œuvre pour pallier les nombreux effets pervers de cette réforme ? Quelle latitude les préfets auront ils pour utiliser leur droit de proposition afin de « rattraper » les communes qui n’auraient pas dû sortir du classement ? Envisagez vous la mise en place d’un moratoire ? La parole

plus zonées. Ces communes étaient maintenues artificiellement depuis 2015 dans le zonage, parce que les gouvernements successifs n’avaient pas souhaité acter la sortie des communes qui ne répondaient plus aux critères.

illisible et peu efficace. En effet, seulement 7 % des communes zonées, depuis 2015, se saisissaient du dispositif. Cette réforme est plus juste grâce à l’actualisation des critères et à la prise en compte des problématiques spécifiques de certains territoires : les territoires de montagne, comme vous le savez, et des départements entiers en déprise déprise démographique continue. Cette réforme est plus efficace grâce au renforcement des exonérations – je veux saluer le travail fait par la sénatrice Espagnac et le sénateur Delcros sur ce sujet. Elle permet de zoner 17 700 communes,

leur expliquer les raisons de la sortie du zonage, et non pas, comme le disait Coluche avec une pointe d’humour, pour leur expliquer comment s’en passer.

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République, de demander au Sénat l’inscription dans notre Constitution de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Oui, j’ai l’honneur de venir devant vous, pour la troisième fois en moins d’un an et demi, afin de vous présenter un texte de compromis, qui, sans rogner sur l’ambition qui est la nôtre, apporte les garanties juridiques indispensables à l’œuvre du constituant. J’espère sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette fois ci sera la bonne, car ce projet de loi, une fois n’est pas coutume, a été précédé de longs travaux parlementaires, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Des votes ont eu lieu, dans des versions différentes, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le texte, très largement adopté à l’Assemblée nationale, arrive désormais devant le Sénat. Vous l’aurez compris, non pas d’une création de la Chancellerie, mais bel et bien d’une proposition de compromis, qui reprend quasi intégralement la version votée par la chambre haute. Si je parle de « compromis », c’est parce qu’une loi constitutionnelle, plus que toutes les autres, doit se concevoir dans une logique de dialogue et de coconstruction. Voter une révision constitutionnelle, ce n’est pas voter la version de l’Assemblée nationale ou rien. Ce n’est pas non plus voter la version du Sénat ou rien. Voter une révision constitutionnelle, c’est faire converger les chambres, car elles disposent toutes deux d’un droit de veto. C’est pourquoi j’ai souhaité que le texte que je vous propose parte de la version votée par le Sénat et, surtout, en respecte les lignes fondamentales, en particulier sur l’encadrement de sa portée. Les Françaises et les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l’attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France. J’ai toujours eu pour le Sénat

Mon état d’esprit est celui d’un garde des sceaux déterminé à convaincre, mais avant tout respectueux des consciences de toutes et de tous dans cet hémicycle. J’en viens aux raisons qui m’amènent aujourd’hui devant vous, et je veux m’arrêter sur la nécessité de cette réforme. Cette nécessité est d’abord J’entends qu’un certain nombre d’entre vous ne souhaitent pas importer des débats venus d’outre Atlantique. Mesdames, messieurs les sénateurs, nul besoin d’aller si loin ! européens – polonais ou hongrois – devraient suffire à vous convaincre. Je rappelle que, alors que l’extrême droite était au pouvoir, voilà encore quelques mois, les Polonaises ne pouvaient avorter qu’en cas de viol ou d’inceste ou quand leur vie était en danger. Il a fallu qu’un parti modéré revienne – heureusement ! – au pouvoir pour que l’espoir renaisse enfin quant au rétablissement de cette liberté de la femme. En Hongrie, les femmes qui souhaitent avorter sont forcées d’écouter au préalable les battements de cœur du fœtus qu’elles portent. Elles attendent toujours qu’une future majorité mette un terme à leur calvaire. Ces parenthèses insupportables dans les droits des femmes, qui sont au mieux des éclipses, au pire des nuits profondes, voilà précisément ce que nous voulons empêcher grâce à cette révision constitutionnelle.

mais bel et bien en France, sur une chaîne française, qu’avant hier encore on associait le nombre d’avortements à celui de morts du cancer et de décès liés au tabac.

Certains affirment que l’IVG ne serait pas menacée. Tant mieux s’ils ont raison, mais, si l’avenir leur donnait tort, mesdames, messieurs les sénateurs, il serait trop tard la République Jacques Chirac a proposé la constitutionnalisation de l’abolition de la peine de mort, cette dernière était elle menacée ? J’ai entendu le président Larcher dire que la Constitution ne devait pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Je respecte son point de vue,… Encore heureux ! … même si – le président Larcher, j’en suis sûr, me le concédera – le principe d’une Constitution est aussi de réunir l’ensemble des droits et libertés fondamentaux,

La liberté de recourir à l’IVG n’est pas une liberté comme les autres, car elle permet aux femmes de décider de leur avenir. Une démocratie ne peut maîtriser pleinement son destin si les femmes qui y vivent n’ont pas la liberté de maîtriser le leur. J’en viens maintenant à la nécessité à la nécessité juridique de cette révision. Disons les choses clairement. Trois principes sont en débat aujourd’hui : la liberté de la femme de recourir à une IVG, la liberté de conscience – en l’occurrence, des médecins et des sages femmes –, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, à l’occasion de sa décision du 27 juillet 1994.

de conscience, donc celle des médecins et des sages femmes, a été reconnue expressément par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision du 27 juin 2001. Cette liberté de conscience a donc, elle aussi, valeur constitutionnelle.

est simplement rattachée à la liberté de l’article 2 de la Déclaration de 1789, sans qu’elle soit d’aucune manière manière consacrée comme un quelconque principe à valeur constitutionnelle ou principe fondamental reconnu par les lois de la République. L’objectif de ce projet de loi est donc de protéger l’IVG dans notre Constitution. rien n’empêcherait une majorité, au Parlement, de contraindre excessivement, drastiquement, cette liberté des femmes ou, pis encore, de l’abolir. s’il est nécessaire d’agir, il faut le faire de manière calibrée, prudente, soupesée. Que les choses soient très claires : le Gouvernement n’entend pas créer un droit absolu, sans limites, opposable. Il s’agit aujourd’hui de protéger cette liberté de la femme, pas de l’étendre. Pour dire les choses plus simplement encore, le Gouvernement veut éviter qu’une majorité future puisse mettre à mal la liberté des femmes de disposer de leur corps. Pour ce faire, le projet de loi reprend – je l’ai dit – une rédaction très proche de celle qui a été adoptée par le Sénat voilà un an.

est à 95 % celui du Sénat. Je réitère ce propos aujourd’hui devant vous. Jugez en par vous mêmes,

cette rédaction accorde, tout comme l’avait fait le Sénat, une place centrale à la loi pour déterminer les conditions d’exercice de cette liberté, et préserve ainsi le rôle le rôle du Parlement pour assortir cette liberté de conditions qu’il estime appropriées. Enfin, contrairement à ce qu’avait voté l’Assemblée le Gouvernement s’est rangé derrière le choix, opéré par le Sénat, de définir le recours à l’interruption volontaire de grossesse comme une liberté. veux m’arrêter un instant, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un point, dont je sais qu’il suscite des débats parmi vous, à savoir le mot « garantie ». Je veux vous rassurer tout de suite – je le dis en particulier au sénateur Philippe Bas – : ce terme ne devrait pas vous inquiéter, car, contrairement à ce que j’ai pu entendre, il ne crée en aucune manière un droit opposable. Par ce mot, le Gouvernement entend préciser l’intention qui guide la plume du constituant, car il ne faut pas perdre de vue que le texte emporte modification de l’article 34 de la Constitution, exactement comme vous l’avez voulu. Or nous savons que l’article 34 de la Constitution est avant tout un article de procédure, dédié à la compétence du législateur. Le terme « garantie » permet de rendre clair

de sa compétence dans le sens de la protection de cette liberté, notamment contre des tentatives législatives de la restreindre drastiquement. le Gouvernement souhaite, en l’inscrivant dans la Constitution, protéger la liberté de recourir à l’IVG, et non l’étendre. D’ailleurs, dans son avis, le Conseil d’État confirme de manière limpide cette position qui est la nôtre : « Par elle même, l’inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le Gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous tend la liberté des médecins et sages femmes de ne pas pratiquer une ainsi que la liberté d’expression. » Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux m’adresser à ceux qui évoquent un « ovni juridique » au sujet de la « liberté garantie ». Je veux, là aussi, les rassurer pleinement : il suffit de reprendre l’article 61 1 de la Constitution, qui renvoie déjà aux droits et libertés que la Constitution garantit ». L’article 13 évoque également « la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation Enfin, dans le titre XII, si cher au Sénat, les articles 72 et 73 évoquent même le cas de « droits constitutionnellement garantis ». Ce terme « garantie », vous le voyez, n’a rien d’incongru. Le texte est clair, tout comme son intention. Qu’il me soit permis de prendre un exemple : même après l’adoption de la présente révision une loi qui viendrait porter à huit mois et demi de grossesse le délai maximal pour pratiquer une IVG serait censurée.

Au reste, mesdames, messieurs les sénateurs, si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est bien pour débattre d’une révision de notre Constitution, et non pour voter je ne sais quelle mesure nouvelle relevant du périmètre du ministère de la santé. Bien sûr, le Gouvernement n’ignore pas les difficultés matérielles et concrètes qui peuvent encore exister dans l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, notamment sur certaines parties du territoire. Mais il s’agit là d’un autre sujet, qui n’est pas d’ordre constitutionnel et qui ne relève pas du périmètre du ministère de la justice. Le Sénat a déjà dit « oui à une protection dans notre Constitution de cette liberté, et je veux saluer ici l’engagement de la sénatrice Vogel. Je veux aussi remercier toutes les sénatrices tous les sénateurs qui, dans chaque groupe politique, au delà des clivages partisans, ont œuvré dans l’ombre du Palais du Luxembourg pour convaincre leurs collègues que, non, ce texte de compromis n’a pas d’effets de bord, et que, oui,

Si le Sénat ouvre, cet après midi, la voie à un Congrès, ce sera en grande partie grâce à vous toutes et à vous tous. Je veux également saluer l’engagement du sénateur Bas, même si je sais, monsieur le sénateur, que vous préférerez toujours votre version à celle du Gouvernement. Cependant, je suis sûr que vous savez, dans votre for intérieur, que le Gouvernement, dans sa version de compromis, a largement repris votre proposition, qui avait permis – il faut s’en souvenir – un premier vote historique il y a un an. Enfin, je veux saluer le travail de la commission et de sa rapporteur, qui, après ne pas s’être opposée au texte lors de son passage en commission, a émis des avis défavorables sur tous les amendements qui seront proposés. Enfin, je souhaite vous faire une confidence je ne serai jamais le procureur du procès en ringardise que certains veulent instruire contre le Sénat.

sans portée juridique, mais des points majeurs, comme le caractère provisoire de la loi, que le Sénat souhaitait souhaitait supprimer, et le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale, que le Sénat avait ajouté dans la loi, contre l’avis du gouvernement

où chaque sénateur doit prendre ses responsabilités, décider en son âme et conscience » : c’est en ces termes que le sénateur Jean Mézard, rapporteur de la loi Veil, concluait son propos liminaire, avant que Simone Veil ne lui réponde, dans son discours Cette responsabilité est aujourd’hui particulièrement lourde. Mais je sais que la nation peut compter sur le Sénat pour délibérer et se prononcer avec humanité, sagesse et sérénité. » Mesdames, messieurs les sénateurs, je fais miens ses mots, et je vous appelle à adopter conforme ce projet de loi constitutionnelle, pour qu’ensemble nous fassions de la France le premier pays au monde à protéger dans sa Constitution la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mesdames, Mesdames, messieurs les sénateurs, et si nous adoptions ensemble ce texte

nous voici réunis pour la troisième fois en moins de seize mois pour examiner l’inscription dans la Constitution de l’interruption volontaire de grossesse. Légalisé depuis 1975, grâce à l’engagement fort de Simone Veil, le droit de recourir à l’IVG est reconnu aujourd’hui comme une liberté fondamentale de la femme. Près de cinquante ans plus tard, le débat qui nous anime n’est pas de savoir si nous sommes favorables ou non à l’IVG : la question est tranchée. Le consensus politique et démocratique est extrêmement clair sur notre attachement à cette liberté fondamentale, non remise en cause aujourd’hui en France. Près de cinquante ans plus tard, la question posée est faut il modifier la Constitution pour inscrire à son article 34 que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une

élargissement aux sages femmes de la possibilité de les pratiquer, remboursement à 100 %, suppression du délai obligatoire de réflexion et du consentement d’un adulte pour les mineurs. Malgré tout, des difficultés persistent. L’accès à un centre de santé sexuelle, le développement de l’éducation auprès des jeunes, la faible valorisation des actes médicaux restent des freins connus. la commission des affaires sociales a confié à notre collègue Alain Milon une mission de contrôle destinée à évaluer la mise en application des lois IVG sur l’ensemble du territoire français. Les réformes nécessaires relèveront de la loi ou du règlement, non de la Constitution.

Or l’inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l’avortement ne saurait se faire en réaction à l’importation d’un débat étranger,… Très bien ! … qui, de plus, n’est pas transposable en France. Cependant, nous ne devons pas rester sourds à ce qui se passe dans d’autres pays, notamment européens. L’ensemble des 27 pays de l’Union européenne autorisent désormais l’IVG. Dans 24 pays, l’avortement est autorisé sous conditions – proches de celles qui existent en France. Seuls deux pays, Malte et la Pologne, fixent des conditions très restrictives, et la Hongrie a imposé, en 2022, l’obligation pour la femme souhaitant avorter d’écouter les battements de cœur du fœtus. Dans le reste du monde, la situation est plus contrastée. L’avortement est autorisé dans seulement 77 pays et complètement interdit dans 22. Mais aucun État ne fait explicitement référence à l’IVG dans sa Constitution, sauf pour l’interdire. Aujourd’hui, aucune contestation du droit à l’IVG n’est portée en France dans le débat politique, comme le reconnaît le Gouvernement dans l’exposé de ses motifs. Aucun parti politique, aucun groupe parlementaire ne s’oppose à cette liberté fondamentale. Le vote massif et transpartisan intervenu à l’Assemblée nationale en faveur de la constitutionnalisation en est la preuve. Toutefois, les effets juridiques de cette constitutionnalisation seront plus que limités. Cette inscription ne sera qu’une consécration constitutionnelle symbolique, comme l’affirme le Conseil d’État dans son avis du 7 décembre dernier. L’inscription noir sur blanc dans la Constitution permettra de consacrer la liberté de recourir à l’IVG, qui acquerra une place éminente dans l’ordre juridique, mais celle ci ne sera nullement sanctuarisée. Certes, sa suppression nécessitera une révision constitutionnelle. Mais notre loi fondamentale a déjà été révisée 24 fois, et un changement de régime n’est jamais impossible La consécration constitutionnelle n’apportera donc aucune garantie juridique absolue, et encore moins une protection renforcée. Depuis 1975, le Conseil constitutionnel a toujours protégé avec force et constance le droit à l’avortement en France. Dans leur décision du 27 juin 2001, les juges constitutionnels ont clairement affirmé que la liberté de recourir à l’IVG était une composante de la liberté de la femme découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel dispose d’ores et déjà de tous les outils juridiques pour protéger cette liberté fondamentale et assurer sa conciliation avec les autres libertés que sont la sauvegarde de la dignité humaine et la liberté de conscience des médecins. La rédaction proposée par le Gouvernement conforte, à notre avis, la recherche d’une simple consécration symbolique dans la Constitution. Proche de la formulation adoptée par le Sénat en février 2023, de loi reprend l’inscription de la liberté de recourir à l’IVG à l’article 34 de la Constitution. De l’aveu même des nombreux constitutionnalistes auditionnés, aucune place dans la Constitution de 1958 ne permet d’accueillir naturellement le droit à l’IVG.

L’inscription à l’article 34 est donc un moindre mal. Cet article procédural énumère les matières qui sont du domaine de la loi. Le législateur étant déjà compétent pour fixer les règles concernant les garanties apportées aux libertés fondamentales, dont fait partie l’IVG,

Cependant, deux différences notables subsistent. La première doit pouvoir être traitée facilement, puisqu’elle porte sur l’utilisation du terme « IVG », au lieu de l’expression « mettre fin à sa grossesse Cette substitution n’est pas neutre : nous savons qu’elle est essentielle pour les défenseurs de la constitutionnalisation symbolique de la liberté de recourir à l’IVG, car c’est le terme de la loi Veil. C’est pourquoi je proposerai au Sénat d’accepter d’inscrire le terme « IVG » dans la Constitution. La seconde soulève plus d’interrogations, puisqu’elle introduit un nouveau concept de « liberté garantie », dont les contours juridiques sont mal définis.

toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet article socle affirme clairement que, dès lors qu’elle est inscrite dans la Constitution, une liberté est garantie. Pourquoi donc le réaffirmer pour l’IVG, et non pour toutes les autres libertés fondamentales ? Pourquoi ajouter cet adjectif redondant, qui alourdit la rédaction de notre Constitution, sans renforcer la portée de ses dispositions ?

Rien n’est moins sûr, car le Conseil constitutionnel ne s’estime lié ni par les avis du Conseil d’État ni par les débats parlementaires. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, la commission des lois du Sénat est favorable à la constitutionnalisation de la liberté de recourir à l’IVG. La défense de cette liberté fondamentale est un combat livré par de nombreuses femmes et de nombreux hommes. Nous devons continuer à agir pour que toutes les femmes puissent accéder à cette liberté sur tout le territoire français, en s’assurant qu’aucune régression ne vienne en limiter les effets. Mais, aujourd’hui, nous sommes avant tout constituant. Le texte que vous allez voter, mes chers collègues, n’est pas une simple loi ordinaire : c’est un projet de loi constitutionnelle. Il définira les termes qui seront inscrits dans notre loi fondamentale. Notre responsabilité est grande Proche du texte adopté par le Sénat en février 2023, ce projet de loi constitutionnelle ne modifie pas fondamentalement les équilibres juridiques. C’est avant tout une avancée symbolique. la commission des lois a considéré que les incertitudes rédactionnelles ne pouvaient retarder l’adoption d’un texte conforme.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à la réflexion, je vous le concède, la gauche a raison : aujourd’hui, en France, la loi Veil est menacée. Le respect de tout être humain dès le commencement de la vie », garanti par l’article 1 de la loi Veil, est menacé, tout autant que la clause de conscience des professionnels de santé et la liberté d’expression et de communication à ce sujet. Simone Veil, de son Panthéon, nous le dit encore, comme elle nous le disait avec toute sa conviction : « L’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue. Vous voudriez faire d’une dérogation un accomplissement, d’une exception un droit absolu et sans limites, d’une réserve un monument. Vous voulez « panthéoniser » l’avortement Mais, dans la Constitution comme au Panthéon, la place est limitée. Et, s’il ne faut toucher à la loi « que d’une main tremblante », il ne faut réviser la Constitution qu’avec la crainte de l’architecte qui touche à la clé de voûte de l’édifice national. Vous voulez panthéoniser l’avortement aux côtés du principe de précaution de 2004, de la garantie des « droits inaliénables et sacrés » de tout être humain de 1946, de la « liberté de conscience » de 1789. Vous voulez faire entrer l’avortement au panthéon des institutions, alors qu’un certain Schœlcher est entré au panthéon des hommes pour avoir mis fin à l’esclavage, qui était pour lui « un attentat contre la dignité humaine ». Au même titre que nous l’avons fait pour les esclaves dans le passé, nous serions bien avisés de réfléchir à l’obtention de la personnalité juridique pour les vies à naître Tenez vous vraiment, mes chers collègues, à rejoindre le dictateur communiste Tito, qui fut le seul dans l’histoire du monde à graver l’avortement dans le marbre d’une constitution, la constitution yougoslave ? « Constituer » signifie « bâtir », « édifier », et ne peut rimer avec « avorter » Chers collègues de gauche, vous n’acceptez pas d’avoir été dépossédés, en 1975, par une élue de droite, soutenue par un gouvernement de droite, de ce qui n’aurait jamais dû quitter ce qui n’aurait jamais dû quitter votre giron idéologique. Cessez de surjouer à vous faire peur et de vous rêver en résistants ! Vous êtes cinglé ! Il n’y a aucune menace sur le droit à l’IVG dans notre pays. Aucune ! Chers collègues macronistes, vous voudriez une victoire symbolique, avec les idées de la gauche et les voix de la droite, pour faire oublier que, du Salon de l’agriculture aux salons de l’Élysée, c’est le désastre permanent pour votre champion ! Le Jupiter de pacotille persiste néanmoins dans son mépris des institutions, en ayant déjà livré la date du Congrès. Chers collègues du Rassemblement national, n’oubliez pas les propos pas si lointains de votre présidente sur la dérive que constituent – je la cite – les « avortements de confort » ! De la dédiabolisation au reniement, il n’y a qu’un pas. L’abandon ne mène jamais à la victoire. Chers collègues du centre et de droite, ne cédez pas à ce qui n’est qu’une opération d’agit prop de la gauche ni à son chantage

Mes chers collègues, je souhaite que nos débats conservent la sérénité qui est la marque de fabrique de notre assemblée… Pas de la gauche ! … et qui contribue à la bonne image de nos travaux. Je n’hésiterai pas, pour maintenir cette sérénité, à faire usage des prérogatives du règlement qui sont conférées à la présidence de séance. Ce rappel étant fait, nous reprenons le cours normal de la discussion.

toute sa société, par la voix de son Parlement, donne tort à M. Ravier et à ses amis ; que notre pays choisit aujourd’hui définitivement son camp ; que la République ne sera plus jamais fragile

Il me paraît fondamental d’inscrire la liberté de recourir à l’IVG dans la Constitution, car il sera beaucoup plus difficile de modifier celle ci que de changer la loi. Monsieur le sénateur Ravier, à votre corps défendant,

! Si j’entends certains arguments juridiques – pas tous –, je pense que la Constitution est au cœur de notre pacte social. Il s’agit également d’y inscrire des principes fondamentaux. fondamentaux. En effet, aucun pays n’est jamais à l’abri d’une majorité politique susceptible d’abroger les dispositions autorisant l’avortement, la liberté d’y recourir et la contraception, ou d’en restreindre l’accès. Je veux saluer ici toutes celles et tous ceux, sur toutes nos travées, qui se sont battus, depuis des décennies comme ces dernières années, pour protéger ce droit. Je pense en particulier à Mme Vogel. Je veux aussi saluer toutes celles et tous ceux qui rendent ce droit effectif dans nos établissements de santé et font de la prévention et de l’accompagnement. Le groupe RDPI se prononcera contre cette motion. Monsieur Ravier, la reconquête de nos droits commence maintenant

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le débat du jour éveille en nous nombre de considérations politiques, philosophiques et morales. À ce titre, ce serait un manque de respect pour chacun d’entre nous que de tomber dans le manichéisme et la facilité.

mais je rappelle que la Constitution est ce que le peuple et ses représentants veulent en faire. Sinon, on pourrait adresser le même reproche à l’intégration de normes complémentaires dans le bloc de constitutionnalité depuis des décennies, jusqu’à remettre en cause celle de la Charte de l’environnement, ce qui ne viendrait à l’esprit de personne. Mes chers collègues, il est vrai de dire qu’aucune formation politique qui concourt régulièrement aux élections ne propose de restreindre l’accès à l’interruption volontaire de grossesse telle qu’elle est permise aujourd’hui et que, à ce titre, aucune menace ne pèserait actuellement sur ce droit acquis pour les femmes. aucune formation politique – j’y insiste – ne menace ce droit, une autre menace persiste à nos yeux : il s’agit évidemment de l’accentuation des revendications politico religieuses, fondamentalistes et communautaristes et du péril islamiste, qui, insidieusement, mène chaque jour une conquête culturelle, politique et fatalement sociétale. observe déjà que d’aucuns de nos compatriotes ne peuvent assumer leur homosexualité dans certains quartiers confisqués, que nos compatriotes de confession juive y sont menacés, que les femmes y sont tenues d’obéir pour préserver leur intégrité physique, quand bien même on leur demande de paraître libres et consentantes. Je crains qu’un jour la faiblesse, la complicité politique et les réalités démographiques n’amènent à des accommodements raisonnables, comme il en existe dans les pays anglo saxons, et que l’on n’en arrive à plusieurs niveaux de droits sur le territoire français. D’un autre côté, c’est le paradoxe des luttes intersectionnelles qui nous menace, celui qui veut nous faire croire que toutes les luttes d’opprimés – réelles ou supposées – convergent et que l’on peut défendre aussi bien les libertés sociétales que la radicalité religieuse. C’est oublier que le principe des intersections est d’être le théâtre de dramatiques collisions ! Non, mes chers collègues, on ne défend pas la liberté de la femme en important, en toute conscience, de nouvelles radicalités conservatrices. Voilà pourquoi je pense, à titre personnel, que nous n’échapperons pas, pour consacrer ce qui constitue aussi notre identité, c’est à dire la liberté de choix et de conscience, à la protection supralégale de nos libertés. Mes chers collègues, je ne crois pas que ceux qui s’opposeront ce jour à cette proposition soient favorables à une restriction du droit à l’IVG, et je m’abstiendrai de tout jugement intellectuel et moral, mais, vous le savez tout comme moi, l’époque ne se prête plus à la nuance ni aux circonvolutions, si entendables soient elles. Pour ces raisons, et dans le respect de la liberté de vote et de conscience de chacun, à titre personnel et comme l’ont fait la majorité de mes collègues du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, je voterai pour l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. La parole

après sa reconnaissance, cette liberté semble fermement ancrée dans notre droit, protégée, et non menacée. Cependant, au delà de la France, cette liberté n’existe pas dans bon nombre de pays. Nous observons, en outre, des reculs au sein de démocraties, y compris en Europe. La Cour suprême des États Unis a elle même rendu, en 2022, un arrêt permettant aux États fédérés de revenir sur cette liberté des femmes. Nous ne pouvons que comprendre l’émotion suscitée par cette décision.

Comme tous les parlementaires, nous avons à cœur de l’encadrer au mieux et de rendre son exercice accessible, chaque fois que cela est nécessaire. Le projet de loi que nous examinons est l’une des initiatives visant à inscrire l’IVG dans la Constitution pour lui donner une protection supérieure à celle que lui confère la loi.

Le cadre légal doit être la seule borne de cette liberté. Si l’IVG figure actuellement dans la loi, sa protection est supralégale. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté d’avorter était l’une des composantes de la liberté de l’individu, ainsi bénéficier l’IVG d’une reconnaissance de valeur constitutionnelle. Une telle reconnaissance n’est toutefois pas gravée dans le marbre, dans la mesure où le Conseil constitutionnel pourrait modifier sa jurisprudence, tout comme la Cour suprême américaine a modifié la sienne.

Rappelons nous l’importance du choix des mots en droit, singulièrement lorsqu’il s’agit de la Constitution. L’IVG, comme toutes les libertés, ne saurait être une liberté absolue. Il est essentiel qu’elle continue à être encadrée par la loi, tant en ce qui concerne les praticiens habilités à la réaliser que s’agissant des délais dans lesquels elle peut être pratiquée. Nous voulons aussi réaffirmer ici notre attachement à la préservation de la clause de conscience des médecins

de souligner que le fait d’avoir choisi la liberté plutôt que le droit est une formulation qui préserve au mieux les équilibres du régime actuel. Nous sommes également attachés à la précision selon laquelle l’IVG est une liberté, et non un droit opposable. Nous considérons qu’il revient au législateur, et non au juge, d’en définir les contours. Nous estimons, à cet égard, que le terme de « liberté garantie » est une formule superfétatoire. La garantie de cette liberté réside bien davantage dans l’inscription au sein de la Constitution que dans cet adjectif déclaratoire. Cela étant,

près de cinquante ans après l’adoption de la loi Veil, nous sommes ici réunis pour écrire un nouveau chapitre dans l’histoire des droits des femmes. Je ne reviendrai pas sur les arguments techniques et juridiques autour de la constitutionnalisation de l’IVG,

L’histoire récente nous a montré que des démocraties libérales, même bien établies, pouvaient revenir en arrière. Nous courons le même risque, car, si le pire n’est jamais certain, le meilleur ne l’est pas non plus. De fait, des réseaux militants, bien organisés et de mieux en mieux financés, s’activent pour remettre en cause ce droit, avec des méthodes de plus en plus pernicieuses. Certaines plateformes vont jusqu’à créer des numéros verts afin de se faire passer pour des organismes publics et dissuader les femmes qui les appellent. Ce n’est pas aux États Unis que ces

la récente affaire CNews, qui a assimilé l’IVG à la première cause de mortalité dans le monde, aux côtés du tabac et du cancer, a eu lieu. C’est en France

Ne péchons pas par excès de naïveté. La France aussi est perméable à ces manœuvres, et, si le droit à l’avortement est encore solidement ancré dans l’opinion publique, il est de notre responsabilité de législateurs de le protéger. évidemment, ce qui compte est aussi l’effectivité de l’exercice de cette liberté : c’est une chose d’inscrire un droit à l’avortement, c’en est une autre d’en garantir le plein exercice.

Je suis d’ailleurs convaincue que ceux qui, un jour, voudront s’attaquer à cette liberté en France ne s’y opposeront pas frontalement et le feront en en compliquant petit à petit l’accès, en restreignant son champ d’application, jusqu’à en faire une coquille vide. L’enjeu aujourd’hui faire en sorte qu’il ne soit pas possible de modifier la loi afin d’interdire le recours à l’interruption volontaire de grossesse ou d’en restreindre les conditions d’exercice au point qu’elle se verrait privée de toute portée. Ne l’oublions pas, partout où l’IVG est interdite, la contraception l’est aussi. De fait, ne nous y trompons pas, derrière le militantisme anti IVG, l’idée n’est pas de nous éviter un acte chirurgical : il s’agit bien de contrôler nos corps de femmes. Constitutionnaliser, c’est envoyer un message à la société d’aujourd’hui comme à celle de demain. C’est affirmer que la reconnaissance solennelle par la République de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, c’est à dire de la liberté de la femme de disposer de son corps, est non pas un simple droit social ou sociétal, mais bien une liberté fondamentale, qui mérite d’être garantie au cœur même de son texte le plus sacré. La Constitution ne doit pas se résumer à un catalogue de procédures institutionnelles. Elle doit traduire la société dans laquelle nous choisissons de vivre, valeurs. Mes chers collègues, certains parmi vous pensent que cette constitutionnalisation est avant tout symbolique. Si tout cela n’est que symbolique, votons ! Nous n’avons rien à perdre. Et si, comme moi, vous pensez que cela protège un peu plus les femmes, votons ! Nous avons tout à gagner.

pendant des siècles, des femmes ont été maltraitées, insultées, condamnées en France parce qu’elles avaient exercé une liberté, inhérente à la condition humaine : celle de choisir leur vie. Pendant des siècles, des femmes ont comparu en France, devant des tribunaux d’hommes, parce qu’elles avaient décidé de disposer de leurs corps. Pendant des siècles, des femmes, qui n’avaient pas les ressources, pas les contacts, sont mortes, en France, des suites d’avortements clandestins, mortes parce que femmes dans une société qui avait décidé que les femmes ne pouvaient être ni libres ni responsables. Depuis le manifeste des 343,

qu’elles demeurent à la merci du bon vouloir du législateur, qui, un jour peut être, les rappellera à la barre ? Ou leur dirons nous qu’elles sont à jamais libres ? Voilà la seule question qui nous est posée aujourd’hui.

tellement convaincus, tellement sûrs de ne jamais vouloir le faire que nous choisissons aujourd’hui de renoncer démocratiquement à la possibilité même de le faire, car nous pensons que cette possibilité ne devrait plus exister en France, de la même manière que n’existe pas, grâce à la Constitution, de réduire de toute portée la liberté de conscience, la liberté d’association ou la liberté d’expression. Ni plus ni moins

que l’IVG est non pas une concession que le législateur a faite un jour et pourrait reprendre un autre, mais un droit, que le législateur avait confisqué et qu’il a fini par rendre à ces femmes qui se sont tant battues pour le reprendre. Je m’adresse aux héritières et aux héritiers de cette droite et de ce centre qui ont voté pour la loi Veil. Si, un jour, une loi menace l’IVG en France et si, ce jour, la Constitution ne peut rien pour l’empêcher, que direz vous, chers collègues, à vos filles, à vos petites filles et à vos nièces ? Pourrez vous les regarder dans les yeux ? Que leur répondrez vous quand elles vous demanderont pourquoi, quand vous en aviez la possibilité, vous avez refusé de les protéger ? Leur direz vous que ce texte contenait le terme « garantie » ? Que la date du Congrès avait été annoncée trop tôt ? Le 20 décembre 1974, la moitié des sénateurs de la droite et du centre ont voté pour la loi Veil. C’était plus qu’à l’Assemblée nationale. Le Sénat comptait sept femmes : cinq de gauche et deux de droite. Toutes ont voté pour Quel message enverrons nous, cinquante ans plus tard, si plus de la moitié d’entre nous vote pour conserver la possibilité d’attaquer un jour la loi Veil ? Chaque voix contre, chaque voix en faveur du droit à la régression sera la démonstration empirique que, oui, l’IVG doit entrer dans la Constitution Je me suis lancée, il y a plus d’un an, avec toutes ces femmes qui ont su montrer, sur ce sujet, ce qu’était faire de la politique en grand, en vrai, pour l’intérêt général – je pense à Laurence Rossignol, Aurore Bergé, Mathilde Panot, Laurence Cohen, Dominique Vérien,

pays tant qu’il en était temps ! Eh bien, aujourd’hui, en France, il est temps. Il est temps d’être au rendez vous de notre histoire, de répondre aux immenses espoirs que nous avons soulevés dans le monde. Aujourd’hui, des Polonaises, des Hongroises, des Américaines, des Iraniennes, des Argentines regardent avec admiration la France s’apprêter à énoncer, sans ambiguïté, que le droit à l’avortement n’est pas sous droit. C’est un droit fondamental. C’est l’une des conditions des sociétés libres et égalitaires. Dès lors, faisons nous à nous mêmes, aujourd’hui, cette magnifique promesse : plus jamais les faiseuses d’anges, les cintres, les aiguilles et les mortes ! Disons à nos filles, à nos nièces, à nos petites filles qu’elles sont aujourd’hui et désormais à jamais libres de choisir leur vie

avec ce projet de loi constitutionnelle, nous avons la possibilité d’inscrire le droit à l’avortement dans notre Constitution. Le souhait de notre groupe est que ce texte puisse être voté dans les mêmes termes qu’à l’Assemblée nationale.

Elle l’est, d’abord, en France, parce que des forces rétrogrades n’ont pas renoncé à la remettre en cause et parce que des forces médiatiques s’organisent pour la contester. Je pense moi aussi aux propos monstrueux qui ont été entendus sur une chaîne d’information – ou plus exactement de désinformation – en continu, visant à nous faire croire que l’IVG serait la première cause de mortalité dans le monde.

Veil… Oui, l’IVG est menacée en France. Elle est menacée en Europe, notamment en Pologne. Elle est menacée aux États Unis, où quatorze États l’interdisent aujourd’hui. Qui peut, par conséquent, affirmer que l’IVG ne serait pas menacée ? Qu’entendons nous par ailleurs ? Que notre Constitution n’aurait pas vocation à être un catalogue de droits sociaux. Il y a là une conception de la Constitution que nous ne partageons pas. Cette conception, au fond, vise à nous faire croire que la Constitution serait un objet juridique froid, qui se limiterait à l’organisation des pouvoirs politiques. Comment expliquer alors que ceux là mêmes qui développent cet argument ne soient pas avares en propositions de loi constitutionnelle n’ayant rien à voir avec la stricte organisation des pouvoirs

il ne faudrait pas que l’on ait la main plus tremblante quand il s’agit d’ajouter des droits dans notre Constitution que lorsqu’il s’agit d’en retrancher.

pour toutes les femmes à travers le monde qui se battent pour que ce droit soit garanti dans leur pays. D’ailleurs, quand bien même le vote de ce texte n’aurait pour fonction que de dire à ces femmes qui nous regardent et qui n’ont pas accès à ce droit aujourd’hui

depuis la décision rendue par la Cour suprême le 24 juin 2022, plus d’une dizaine d’États américains ont totalement interdit l’avortement, pour la plupart sans aucune exception, même en cas Dans certains États, l’abject s’incarne même, puisque la loi incite les citoyens à lancer des poursuites à l’encontre des femmes soupçonnées d’avoir avorté. En Europe, de la Pologne à l’Italie, en passant par la Hongrie, sous la pression de mouvements dits « pro vie », les conditions de l’accès à l’IVG reculent. Certes, nous ne sommes pas de ces pays, mais nous avons en commun avec ces nations quelques fondements démocratiques. En France, le droit à l’avortement n’est pas à l’abri des conservatismes. Il convient tant de s’en émouvoir que de se tenir en alerte. D’ailleurs, dimanche dernier, une chaîne de télévision privée française exposait une infographie plus que douteuse faisant de l’IVG la première cause de mortalité dans le monde. Plus qu’une maladresse, c’est une manipulation honteuse. Soyons cartésiens : si l’interruption volontaire de grossesse n’était pas directement menacée, pourquoi aurions nous ce débat ? Pourquoi vouloir constitutionnaliser l’IVG ? Sans doute parce que, à ceux qui pensent qu’elle est une évidence, nous devons opposer la prudence, en enfermant dans la loi fondamentale un droit acquis de haute lutte par les femmes et pour les femmes.

J’entends par ci par là que constitutionnaliser l’IVG ne serait que symbolique. Mais quel symbole ! D’ailleurs, le débat n’est pas tout à fait tranché par les constitutionnalistes. Quoi qu’il en soit, la France doit se poser en pays des Lumières et être au rendez vous de l’histoire, comme elle l’a toujours été.

en octobre 2022, la proposition de loi constitutionnelle déposée par notre collègue Mélanie Vogel, que je salue ; puis, en février 2023, un nouveau texte issu de l’Assemblée nationale. C’est notre troisième rendez vous. Il nous oblige

Bas, qui attribuait simplement et efficacement au législateur la charge de déterminer les conditions « dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».

Certes, il est légitime de s’inquiéter du risque d’inflation des droits constitutionnels, qui pourrait affaiblir les droits concernés, mais, là encore, nos éminents constitutionnalistes ne sont pas tous d’accord. Nous entendons l’alerte, et, si nous observions une dérive un jour, il faudrait s’y opposer fermement. s’agit aujourd’hui d’asseoir un droit face à un enjeu sociétal fort. Bientôt cinquantenaire, la loi Veil a vu son cadre légal s’améliorer au fil du temps. Son inscription dans la Constitution n’est que la suite logique d’une avancée fondamentale pour la dignité des femmes. Mes chers collègues, le RDSE espère voir la raison l’emporter, avec un vote conforme du Sénat. Faire un demi choix reviendrait à faire de l’IVG un demi droit. Or les femmes doivent accéder à une liberté pleine et entière, avec, pour seule conscience, la leur. La parole

« Le passé ne meurt jamais. Il ne faut même pas le croire passé », écrivait William Faulkner. Ces mots résonnent avec une acuité particulière aujourd’hui, alors que nous sommes témoins, à l’échelle mondiale, de remises en question des droits des femmes, notamment du droit à l’interruption volontaire de grossesse.

gravant dans le marbre de la loi fondamentale une protection pour toutes les femmes, quel que soit leur milieu, nous garantirons sa résistance à l’épreuve du temps et aux vagues populistes qui pourraient frapper notre pays. chers collègues, je vous le dis avec force : arrêtons de croire naïvement que ce qui se passe chez nos voisins ne pourrait se produire dans notre pays. Cette croyance les attaques envers les droits des femmes à disposer de leur corps, notamment chez ces pays voisins, nous obligent à faire preuve d’une extrême vigilance. Aux États Unis, nous avons été témoins de restrictions sévères et d’interdictions de l’IVG dans quatorze États, marquant un recul dramatique pour les droits des femmes.

La Pologne, sous la dernière majorité gouvernementale, a restreint le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ne rendant celle ci légale qu’en cas de viol ou d’inceste ou lorsque la vie de la mère est menacée.

tel un ultime acte de torture. Ces exemples internationaux nous rappellent la fragilité de nos libertés et la nécessité de les protéger de manière inébranlable.

envisager de laisser place à un quelconque recul sur ce droit équivaut à accepter de mettre en danger des milliers de femmes dans ces régions, dans un futur incertain. Face à ces réalités, la France, en tant que nation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être à l’avant garde. de l’IVG dans notre Constitution n’est pas seulement un acte de protection. Il l’est, bien sûr, mais il s’agit aussi – nous devons l’assumer – d’un acte symbolique, d’un message fort envoyé aux femmes du monde entier, par lequel nous affirmons nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Par là même, notre pays restera, comme il l’a toujours été au travers des siècles, un phare de liberté, un phare en faveur des droits des femmes, un phare en faveur des droits humains. Simone Veil elle même a su porter la voix des femmes, avec force et opiniâtreté, face à l’adversité et au scepticisme. qui nous rassemble – celle pour le droit des femmes à disposer de leur corps –, résonne comme l’aboutissement de près de deux siècles de combats, en écho aux aspirations pour l’égalité exprimées par Olympe de Gouges dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791,

chers collègues, l’histoire récente à travers le monde nous montre que la montée des gouvernements populistes et nationalistes a fréquemment entraîné un resserrement des libertés, affectant particulièrement les droits des minorités et des femmes, qui sont les premiers à être affectés par ces virages idéologiques. À ces populistes et nationalistes de notre pays, qui s’imaginent que débattre de l’IVG serait une perte de temps, que le Parlement et le Gouvernement devraient se pencher sur des sujets « plus importants », je veux répondre que rien n’est plus important que les droits des hommes et des femmes : c’est l’essence même de notre République, qu’ils méprisent tant. À ces populistes et nationalistes de notre pays, je rappelle que les événements qui se sont récemment déroulés dans nos rues, certains documents et courriers que nous recevons ou encore les chaînes d’information en continu qui diffusent des contre vérités témoignent des menaces persistantes et des attaques régulières contre ce droit fondamental. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux façonnent de nouvelles croyances, où près d’un jeune sur dix croit à des théories aussi dépassées que celle selon laquelle la sœurs, aux femmes et aux petites filles de ce pays, je refuse de les imaginer vivre dans la peur, dans un monde où leur corps ne leur appartiendrait pas, où une grossesse non désirée pourrait bouleverser leur destin. Parce qu’aucune femme, en France et dans le monde, ne se réveille un matin en pensant que c’est le jour idéal pour prendre la décision déchirante d’avorter. Parce qu’aucune femme, en France et dans le monde, ne considère l’IVG comme une option de contraception parmi d’autres. Parce qu’aucune femme, en France et dans le monde, ne recourt à l’IVG avec légèreté et insouciance. Parce qu’aucune femme, en France et dans le monde, ne se tient devant cette porte sans se demander si elle pourra la franchir, si elle aura la force de poursuivre. Parce qu’aucune femme, en France et dans le monde, ne doit être réduite à un rôle qu’elle n’a pas choisi, par peur ou par manque de choix. Non, cher collègue, « l’IVG de confort » n’existe pas ! De tels propos sont non seulement réducteurs, mais aussi et surtout insultants pour les femmes. La liberté de choisir, à laquelle nous sommes tous attachés dans cet hémicycle, est, au fond, l’une des libertés sociales les plus fondamentales. Refuser de l’entendre, c’est réduire la femme à un simple utérus et à un rôle reproducteur. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, par devoir et pour l’histoire, pour Simone Veil et pour toutes les femmes qui se sont battues et se battent encore à travers le monde, gravons dans le marbre de notre Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse en France ! La parole

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « Quand je dépose le texte, c’est à la suite d’un événement que j’ai connu comme avocat. Une jeune femme est livrée à une faiseuse d’anges, victime de septicémie, elle meurt, à 18 ans. […] Je trouve cela tellement injuste et je me dis : il n’est pas pensable qu’on ne puisse être maître de son corps, du fruit que l’on porte, et si on ne veut pas de ce fruit, on a le droit de le rejeter, on n’est pas obligé d’être mère. Ces mots sont ceux d’Henri Caillavet. Ils ont été prononcés en 1947, à l’occasion de ce que je pense être la première proposition de loi consacrée à la dépénalisation de grand sénateur, grand humaniste, grand législateur, soit associé aujourd’hui à ceux de Gisèle Halimi, de Simone Veil et d’Yvette Roudy, à qui nous devons la dédiabolisation de l’avortement, la légalisation de l’IVG et son remboursement. Je souhaite, mes chers collègues, répondre à quelques arguments – nous en avons échangé un certain nombre depuis un an et demi – qui me paraissent devoir être sérieusement discutés.

Si nous pensons indispensable de protéger le droit à l’avortement en l’inscrivant au sommet de la hiérarchie des normes, c’est parce que les anti IVG n’ont jamais renoncé depuis la loi Veil. Cela m’amène au deuxième argument

n’y a pas de menace. Et nous le devons d’abord aux Français, qui, à plus de 80 %, soutiennent le droit à l’avortement et l’ensemble des réformes que nous avons conduites pour en favoriser l’accès. Ils sont aujourd’hui le meilleur bouclier, le bouclier citoyen de la protection de l’IVG. Je veux les saluer et les en remercier. Mais il faut voir plus loin, tant dans le temps que dans l’espace. Partout où les extrêmes droites, les ultraconservateurs, les nationaux populistes, les totalitaristes, les illibéraux – quel que soit le nom qu’on leur donne leur donne – ont accédé au pouvoir, l’avortement et les droits des femmes sont leurs cibles. Trump aux États Unis, Bolsonaro au Brésil, Milei en Argentine, Orbán en Hongrie, Meloni en Italie, Droit et justice (PiS) en Pologne, le ministre de la santé de Poutine… Tous ces gens sont les amis de Mme Le Pen : ce sont ceux avec qui elle danse la valse, déjeune, complote ! Ce sont ceux qui la financent. Et tous, sans exception, ont la même obsession : restreindre les droits des femmes à l’IVG, poursuivre les femmes qui y recourent, criminaliser et harceler les militantes et les soignantes qui viennent au secours des femmes. Tous, sans exception ! Je ne crois pas à une quelconque exception de l’extrême droite française, à l’idée d’un microclimat qui nous protégerait. En revanche, je crois à la, et je ne la vois pas uniquement chez les islamistes ! Je la vois aussi chez nous,

Ce soir, puis au Congrès, nous serons fidèles à la grandeur de la France, ce pays précurseur, phare des droits humains, qui éclaire et encourage celles et ceux qui luttent pour leur émancipation.

chers collègues, cinquante ans après son adoption, la loi Veil est largement entrée dans les mœurs. Nous devons cette acceptation sociale à l’équilibre sur lequel elle repose primauté de la liberté de la femme au cours des premières semaines de grossesse, primauté de la protection de l’enfant à naître ensuite. Cet équilibre fondamental a valeur constitutionnelle. En effet, depuis sa décision de 2001, le Conseil constitutionnel vérifie que la loi ne rompt pas « l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Après cinquante années d’application continue d’une loi qui n’est plus contestée et d’un contrôle constitutionnel vigilant, on ne peut pas dire que l’interruption volontaire de grossesse soit en danger Et, si de nombreux problèmes demeurent, ils ne sont pas d’ordre juridique. Aussi n’est ce pas sans circonspection que nous avons vu arriver, depuis quelque temps, des propositions d’inscription d’un droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, avec des rédactions qui n’étaient pas seulement destinées à protéger la loi Veil, mais qui visaient aussi à ouvrir la voie à une rupture de l’équilibre constitutionnel que j’ai décrit, en faisant de l’IVG un droit opposable, absolu, sans limites. Malgré les réserves que m’ont inspirées les premières propositions dont nous avons discuté, j’ai admis, dans son principe, l’idée qu’une sécurité supplémentaire pouvait justifier une mention dans la Constitution – pas n’importe laquelle Cette ouverture a été assortie de conditions simples : que l’équilibre de la loi Veil soit préservé et que l’espace constitutionnel reste reste suffisamment ouvert pour que le législateur puisse y faire évoluer la loi sans remettre en cause cet équilibre. Le Sénat a adopté, l’an dernier, son propre texte, prévoyant que « la loi détermine les conditions » – c’est à dire aussi les limites dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Il a ainsi reconnu une liberté individuelle, et non un droit opposable qui n’aurait à se confronter à aucune autre exigence constitutionnelle. le lot commun de toutes les libertés que d’être limitées par le respect de principes constitutionnels de même force – ici, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, c’est à dire la protection de l’enfant à naître. Tel a été le choix du Sénat. Nous ne devons pas aujourd’hui en altérer la clarté. Ce texte a inspiré la rédaction proposée par le Président de la République. On y retrouve, en effet, deux mots essentiels : « conditions qui indique que la liberté de l’interruption volontaire de grossesse ne peut être sans limites ; « liberté », terme préféré à celui de « droit », pour éviter tout glissement sémantique et juridique vers un droit créance. Deux différences apparaissent cependant entre la proposition de chef de l’État et notre texte. La première consiste à ne plus inscrire « la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse », mais seulement sa « liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » – et non pas, monsieur le garde des sceaux, « la liberté des femmes de disposer de leur corps », comme vous l’avez dit, peut être par approximation de langage… Cette formulation fixe dans la Constitution une terminologie conçue pour ne pas nommer l’avortement dans la loi Veil. J’en prends acte. La seconde différence est beaucoup plus critiquable, car elle créerait une ambiguïté dans le texte constitutionnel : il s’agit du recours au concept étrange de « liberté garantie ». Il y aurait donc, dans la Constitution, des libertés et des droits « garantis », et d’autres qui ne le seraient pas. Une telle hiérarchie entre libertés constitutionnelles laisse songeur. La mission du Conseil constitutionnel sera de rechercher l’effet utile de l’adjectif « garantie », sans faire au constituant l’injure de considérer qu’il aurait pu l’écrire pour ne rien dire. Ne nous y trompons pas : il s’agit, en réalité, de réintroduire, de manière ambiguë, la notion de droit opposable. Mais, en démocratie, c’est à la représentation nationale, et non au juge, de veiller à ce que l’interruption volontaire de grossesse soit accessible à toutes les femmes ! Si l’adjectif « garantie » n’a aucune portée, comme vous le soutenez, monsieur le garde des sceaux, pourquoi l’ajouter ? Par ailleurs, s’il doit en avoir une, il vaut mieux le retirer ! C’est tout le sens de l’amendement que j’ai déposé avec Bruno Retailleau, président de notre groupe, et de nombreux collègues, à l’instar de notre rapporteur. Mes chers collègues, je le dis à chacune et à chacun d’entre vous, y compris à celles et à ceux qui, en conscience, veulent s’opposer à toute inscription constitutionnelle : si cet amendement n’était pas voté, … Il faut conclure. … c’est une version ambiguë de la révision constitutionnelle qui risquerait finalement

de l’article 1 de la loi Veil : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

raisons : ne pas passer pour un militant anti avortement ; privilégier le symbole au droit ; être le relais d’une opinion publique qui serait très favorable à une constitutionnalisation, même partielle, de la loi Veil partielle, de la loi Veil ; être les seuls au monde à inscrire l’interruption volontaire de grossesse dans notre texte fondamental, et prétendre que cela ferait de notre pays l’avant garde du progrès… Permettez moi d’exprimer quelques doutes. Peut on voter ce texte malgré la piètre qualité d’une énième proposition de rédaction de l’article constitutionnel, dont le seul mérite était de mettre d’accord Mathilde Panot et Marine Le Pen à l’Assemblée nationale ? malgré le fait que l’équilibre intrinsèque de la loi de 1975 ne soit absolument pas repris

En cas d’avènement d’un président illibéral, d’un gouvernement illibéral, d’une majorité illibérale, combien de temps faudrait il à ceux ci pour prendre le contrôle politique du Conseil constitutionnel ? Mes chers collègues, rappelons nous la parabole de la paille et de la poutre : ce n’est certainement pas cette inscription constitutionnelle qui répondra à la fermeture de 130 centres IVG qui a eu lieu ces dix dernières années dans notre pays ou qui empêchera CNews de faire des comparaisons stupides ! Le débat de l’accès est le seul qui vaille – je le dis comme membre et même comme militant de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Eh bien ! Mes chers collègues, la volonté de mettre « quelque chose » dans la Constitution ne saurait l’emporter sur le raisonnement juridique le plus simple.

pour tenter de convaincre les derniers indécis, les hésitants sur le sujet qui nous occupe. J’irai donc droit au but.

Il est vrai que la décision américaine a été un électrochoc pour la société française. Comment, dans une démocratie avancée, l’IVG pouvait elle être menacée ?

Il me semble que notre position doit d’abord tenir à l’idée que nous nous faisons du rôle du législateur – pas n’importe quel législateur : le législateur auquel nous demandons de modifier la norme juridique supérieure en droit français

qui empêcherait la liberté des femmes de recourir à l’IVG de s’exercer ? Je ne crois pas. Je crois même à l’inverse que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui figure dans le bloc de constitutionnalité permet de puiser la force constitutionnelle de cette liberté. C’est en tout cas comme cela que le Conseil constitutionnel l’a écrit. Sommes nous en train de clore un débat qui agiterait la société et, en conséquence, notre vie politique sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse ? Je ne crois pas non plus. Bien sûr, il y a encore en France des gens hostiles à l’interruption volontaire de grossesse. Ils ont parfaitement le droit de le penser,… Oui ! … cela s’appelle la liberté d’expression. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec notre collègue Mélanie Vogel : oui, ils ont ils ont perdu la bataille. Nous vivons dans une société qui, majoritairement, reconnaît la légitimité de la liberté des femmes d’avoir accès à l’IVG.

allusion non pas à des faits, assez rares au demeurant, qui se produisent en France, mais bien à la décision de la Cour suprême des États Unis dans un pays où, oui, le débat sociétal sur l’IVG est extrêmement fort. C’est la mondialisation ! Ces textes font aussi référence à des faits qui se passent dans des pays qui sont sans doute proches du nôtre,

Est ce le rôle de la Constitution que d’émettre des symboles ? C’est un symbole de la République ! Est ce le rôle de la Constitution que d’envoyer des signaux au reste de l’humanité ? Pour ma part, je ne le crois pas. Pardonnez moi d’être un peu terre à terre, mais, une fois que nous aurons acquis ce merveilleux symbole,

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est la troisième fois que nous avons à répondre dans cet hémicycle à la question suivante : souhaitons nous inscrire l’interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution ? Il y a un an, ici même, au Sénat, nous y répondions positivement. Depuis, l’Assemblée nationale s’est prononcée à une très large majorité pour approuver ce projet de loi constitutionnelle. Aujourd’hui, une étape importante reste à franchir, celle de concrétiser cette volonté commune en nous accordant sur le texte. Je forme le vœu que nous y parvenions. Le texte constitutionnel qui nous est soumis est le fruit d’un débat parlementaire nourri, engagé depuis plus d’un an. Notre travail législatif aura permis de cheminer collectivement dans l’écoute et le respect des différentes sensibilités. C’est une belle démonstration de la vitalité du débat parlementaire. Je veux ici saluer l’engagement de notre rapporteur Agnès Canayer sur un sujet sensible, complexe, qui touche à l’intime. Je tiens également à saluer la position de la commission des lois, qui a pris acte du texte sans proposer de le modifier. Pour ma part, je crois profondément que le droit à l’IVG a toute sa place dans notre Constitution. Constitution. En effet, notre Constitution est le texte au sommet de notre hiérarchie des normes. Elle consacre des droits et des libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. Elle est aussi le socle des grands principes de notre pays. La Constitution est cet acte fondateur par lequel notre société se constitue une identité et décide de l’ordre sociétal voulu. Le droit à l’IVG y a toute sa place, car il fait partie intégrante de la liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps. La question qui nous est posée est donc finalement assez simple : souhaitons nous inscrire dans notre texte fondamental cette liberté pour les femmes à laquelle nous sommes tous profondément attachés ? Il me semble que le Conseil d’État, au travers de son avis, nous éclaire en affirmant que l’IVG ne fait l’objet d’aucune consécration constitutionnelle en tant que telle. Dès lors, élever ce droit au rang constitutionnel est indéniablement une protection supplémentaire. Si la situation américaine n’est à mon sens pas comparable à la situation française, faut il réellement que pèse une menace pour sécuriser un droit ou une liberté ? Je ne le crois pas. Notre Constitution a cette force de sanctuariser des principes auxquels il ne doit pas pouvoir être dérogé. Sa force, c’est aussi de savoir s’adapter aux évolutions et aux attentes de notre société. Enfin, sa position au sommet de notre ordre juridique est un rempart à d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans le futur. Il suffit pour s’en convaincre de se tourner vers des pays européens comme la Pologne ou la Hongrie. Ces exemples illustrent à quel point la situation peut évoluer défavorablement pour le droit des femmes en général, et le droit à l’avortement en particulier. Alors même que nous pensions tous que ces droits étaient acquis, nous C’est pourquoi, mes chers collègues, il me semble nécessaire de continuer à réaffirmer et à protéger ces droits fondamentaux acquis par des générations de femmes. Ce texte constitutionnel nous livre une rédaction équilibrée, qui reprend quasi intégralement les termes votés ici même au Sénat il y a un an, grâce à l’amendement de notre collègue Philippe Bas. Le terme « garantie » doit s’entendre comme une protection supplémentaire et non comme un droit opposable. C’est notre volonté aujourd’hui de législateur, demain de constituant. En tout état de cause, l’inscription de l’IVG dans la Constitution ne doit pas éluder les difficultés préoccupantes de l’effectivité du droit à l’avortement : cent trente centres IVG ont fermé ces quinze dernières années. Ces chiffres appellent vigilance et action, comme l’a rappelé notre président Gérard Larcher. Ma conviction n’en demeure pas moins

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je me félicite que nous soyons réunis ce soir dans l’espoir de faire aboutir la constitutionnalisation de l’IVG. J’ai la certitude qu’avec le recul nous regarderons cette soirée comme un moment précieux de l’histoire de notre République, tout comme l’inscription dans notre Constitution de l’abolition de la peine de mort en 2007. Si le séisme provoqué par la révocation de l’arrêt aux États Unis a donné toute sa force à cette revendication, soutenue d’ailleurs depuis 2018 par les socialistes, les menaces qui pèsent sur l’IVG n’épargnent pas non plus le continent européen. Je pense notamment à la Pologne où seules les IVG en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère sont autorisées, à la Hongrie où les femmes souhaitant avorter sont obligées d’écouter battre le cœur du fœtus. Au regard de la montée de l’extrême droite dans notre pays, il est illusoire d’imaginer que nous serons éternellement à l’abri de telles régressions. C’est pour cela que nous appelons, tant qu’il est encore possible de le faire, à cette constitutionnalisation qui enverra ce message fort : le droit des femmes à disposer de leur corps est inaliénable. J’espère qu’une telle victoire nous donnera l’impulsion nécessaire pour garantir l’effectivité de ce droit pour toutes les femmes, y compris celles qui vivent en zone rurale. Faute d’offre de soins suffisante, l’accès à l’IVG est en effet marqué aujourd’hui par de fortes inégalités territoriales, qui pénalisent surtout les femmes isolées et les femmes précaires. Rappelons que treize départements ne comptent aucun gynécologue et que 18 % des femmes réalisent leur IVG hors de leur département. « Je me bats pour le droit de la femme à choisir ses maternités », déclarait Gisèle Halimi. Soyons ce soir à la hauteur de cette ambition.

L’injustice est l’hypocrisie patronnée par la morale. » C’est par ces mots que la gynécologue Marie Andrée Lagroua Weill Hallé, tard le Mouvement français pour le planning familial, évoquait l’arrivée à l’hôpital des femmes qui venaient d’avorter clandestinement. Aujourd’hui, soixante ans après et malgré la légalisation de l’avortement qui a suivi, cette phrase résonne toujours dans notre actualité. injustice » est toujours d’actualité, au regard des inégalités d’accès géographiques et sociales à l’IVG sur notre territoire. L’« hypocrisie » est toujours d’actualité, lorsque, d’un côté, il est dit que le droit à l’IVG n’est pas menacé dans notre pays et que, de l’autre, le corps des femmes fait l’objet d’un débat public incessant et redevient soudain l’instrument d’un « réarmement » dit démographique. « Patronnée par la morale », c’est toujours d’actualité, lorsque, voilà quelques jours encore, les femmes étaient accusées d’être à l’origine de la première cause de mortalité dans le monde. Toujours d’actualité, mais peut être plus pour longtemps, si nous décidons aujourd’hui de prendre ce tournant historique en constitutionnalisant l’IVG. En votant aujourd’hui en ce sens, nous commençons à graver dans le marbre de la République « mon corps m’appartient », « notre corps nous appartient ». Cette liberté de choix doit dépasser tous les débats partisans, religieux et individuels. enfin une réalité constitutionnelle, parce que les droits fondamentaux concernent aussi les femmes. « Il suffira d’une crise », disait Simone de Beauvoir. ? Elle aurait pu ajouter : rien n’est jamais acquis pour les femmes. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de faire cesser cette insécurité. Regardons ce qui s’est passé chez nos voisins hongrois et polonais. Oui, l’IVG est un droit précaire qu’il faut protéger. Prenons les devants et protégeons avec force ce droit fondamental. Nous ne savons jamais de quoi les lendemains sont faits. La Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est bien le devoir de la loi fondamentale que de protéger et de garantir les droits les plus fondamentaux. Il est bon et apparemment nécessaire de le rappeler. Si, aujourd’hui, nous œuvrons à la garantie de cette liberté dans la Constitution, demain, nous continuerons à lutter pour que ce droit soit effectif. Quand les moyens manquent, quand les stocks de médicaments sont vides, quand les forces anti avortement s’organisent pour piéger les femmes, quand les services publics de santé sont défaillants, c’est bien l’accès des femmes à ce droit qui est compromis. Si l’inscription dans la Constitution est une avancée nécessaire que nous saluons, il ne faudrait pas la croire suffisante. Disposer de son corps, c’est choisir d’avoir un enfant ou non. Déjà, dans l’histoire, les femmes ont été victimes de la volonté de l’État de contrôler leur corps dans un sens comme dans l’autre. Je ne peux pas m’empêcher de penser à un épisode trop peu connu de l’histoire de mon département, La Réunion. Entre 1960 et 1970, les femmes réunionnaises ont été victimes de la politique antinataliste de l’État français. Les plus fragiles d’entre elles ont subi des stérilisations non consenties et des avortements forcés à l’époque où la loi interdisait l’avortement Les dérives se sont produites, parce que des politiques bien intentionnés prétendaient agir ainsi dans l’intérêt des femmes elles mêmes. En d’autres mots, ils s’étaient affranchis des limites de la loi dont on a parlé tout à l’heure. Et c’est bien pour réaffirmer que le corps des femmes ne doit pas être un espace contrôlé par l’État que nous voterons pour ce projet de loi constitutionnelle. Il faut conclure ! individuelle, première et physique dans la Constitution, c’est admettre que la femme est la mieux placée pour décider pour elle même.

constitutionnelle, je souhaite en souligner l’importance et la gravité, ainsi que l’opportunité qu’il représente. Près de cinquante ans après l’adoption de la loi Veil, le texte que nous examinons prévoit d’élever la liberté des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse au rang constitutionnel. Il s’agit bien d’un moment historique. En conférant à ce choix fondamental la protection suprême de la Constitution, nous réaffirmerions haut et fort que l’IVG et la maîtrise par les femmes de leur fécondité et de leur corps ne relèvent ni d’une tolérance, ni d’une faveur, ni même encore d’une simple exception, mais constituent bien des principes fondamentaux inscrits au plus haut de la hiérarchie des normes. Dans un contexte où le droit à l’avortement est menacé dans de nombreux pays, notre action enverrait un message d’espoir et de soutien aux femmes d’Europe et au delà. Bien que le recours à l’IVG ne soit pas menacé actuellement en France, il est important de rappeler, comme l’a souligné le Conseil d’État, qu’il n’est pas protégé par une disposition de valeur supérieure. Aussi est il vulnérable aux aléas politiques et sociaux. La rédaction de compromis proposée s’inspire largement de celle qui a été adoptée par notre assemblée sur proposition du sénateur Philippe Bas. Son adoption conforme serait un véritable motif de satisfaction pour notre assemblée. il s’agit bien de garantir la liberté des femmes, tout en offrant une certaine flexibilité permettant au législateur d’adapter le cadre juridique entourant l’IVG. l’émancipation des femmes et la protection de leurs droits font souvent l’objet de beaux discours dans notre assemblée. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité historique de joindre le geste à la parole. J’espère sincèrement que notre assemblée saura être à la hauteur de cet enjeu et que la liberté, l’autonomie des femmes, ainsi que le respect de leur corps et de leur droit

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre présence nombreuse montre l’importance que chacun attache au moment politique que nous allons vivre ensemble dans quelques instants. Le débat qui nous anime aujourd’hui est très attendu de la société française et le garde des sceaux a raison de dire que nous sommes regardés ce soir. En effet, quelle que soit notre position, elle est souvent liée à de très fortes convictions. Ma conviction profonde, sincère, est que le droit absolu à disposer de son corps est une condition indispensable à l’existence de toutes les autres libertés. Fruit d’un long combat, c’est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les hommes. Mes chers collègues, partout dans le monde aujourd’hui s’élèvent des voix et des actions pour restreindre et bafouer le droit à l’avortement. Les exemples sont nombreux. À l’échelle internationale, il y a désormais une coalition d’États qui mène d’âpres offensives contre les droits des femmes, donc contre les droits humains. Le climat n’a jamais été aussi inquiétant, cela a été rappelé à plusieurs reprises lors de la discussion générale. Je pourrais citer l’exemple du planning familial de Lille, dont les locaux ont été tagués de propos insultants à l’égard des femmes il y a quelques jours. La constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse permettra d’envoyer un signal fort, tant à l’échelon national qu’à l’échelon international, un signal d’absolue conviction que garantir l’accès à l’IVG est cardinal et d’une importance telle qu’il ne pourra pas être remis en question. Mes chers collègues, je respecte les sensibilités qui se sont exprimées

! Le Gouvernement a enfin pris ses responsabilités. Nous avons un véritable rendez vous avec l’histoire. Ne le manquons pas ce soir Monsieur le président, aujourd’hui, et c’est un moment rare dans la vie parlementaire, nous avons la possibilité de faire l’histoire.

pour la défense de ce droit fondamental. Nous sommes regardés par les Françaises et les Français et nous sommes attendus pour graver dans le marbre de notre Constitution le droit à l’IVG. Près de 90 % de nos compatriotes soutiennent ce texte. Certains ont dit au cours de ce débat

Là bas aussi, des responsables publics avaient prétendu que cela ne serait jamais le cas, qu’il n’était pas nécessaire de placer ce droit au sommet de la hiérarchie des normes juridiques de leur pays,

Devenons le premier pays au monde à constitutionnaliser ce droit fondamental.

par le travail parlementaire des sénatrices de toutes les travées de notre hémicycle. C’est grisant de voir qu’après deux passages au Sénat nous avons aujourd’hui l’occasion de répondre à une demande de protection des Françaises. Il faut le redire : ici, personne ne prend à la légère cette modification de la Constitution. Personne ici ne considère que nous pouvons faire entrer dans la Constitution nos humeurs ou l’air du temps. En revanche, oui, nous voulons aujourd’hui protéger les femmes des vents mauvais qui soufflent ou souffleront à l’avenir sur notre démocratie. Oh… C’est avec humilité que nous allons voter aujourd’hui, parce que nous ne sommes qu’un petit maillon de la chaîne que constitue ce long combat féministe. C’est en remontant cette chaîne, cette longue histoire du combat pour l’égalité des femmes et des hommes, cette longue histoire faite de drames et de luttes menées par nos grands mères, nos mères, nos sœurs, que nous savons à quel point le moment est important et tout ce que nous leur devons. Ce qui rentrera dans la Constitution, c’est la garantie d’une liberté essentielle, celle des femmes à disposer de leur corps. C’est une nouvelle manifestation du grand principe républicain d’égalité. Laissons nous griser par le moment, pour les Françaises et pour toutes celles et tous ceux qui sont attachés à faire vivre nos libertés et nos principes républicains. Votons ce texte conforme. Envoyons ce beau signal à toutes les démocraties aujourd’hui confrontées à la résistance et aux néoconservateurs. Rendez vous lundi à Versailles

la Constitution en 1958, il en a fallu des combats et il en faudra encore. Il a fallu attendre juillet 1965 pour que le Parlement vote une loi autorisant les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom

de nos mères, de nos grands mères, des féministes, des associations, des militantes, des militants qui ont œuvré pour que ce moment puisse avoir lieu

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a des moments historiques qu’il faut savoir sentir et appréhender. Celui qui nous rassemble aujourd’hui appartiendra indéniablement à l’histoire perpétuelle du combat en faveur du droit des femmes. Garantir la liberté de la femme à disposer de son corps se révèle un véritable combat dans le combat, peut être le plus ardu à gagner. Or le Sénat, par sa prudence, son réalisme et sa sagesse – triptyque cher à Alain Poher –, a souvent su être au rendez vous de ces moments historiques. Aujourd’hui, je crois que nous avons précisément besoin de sa prudence, de son réalisme et de sa sagesse. Prudence de garantir aux femmes une protection juridique maximale, en constitutionnalisant la liberté de recourir à l’IVG. Réalisme d’observer que la France n’est pas un pays isolé et que, partout, cette liberté est constamment remise en cause et attaquée, quand elle n’est pas tout simplement niée. Sagesse, enfin, de ne pas insulter l’avenir et d’anticiper, puisque gouverner, c’est prévoir. Certes, la Constitution n’est pas uniquement un catalogue de droits, mais au travers de ces droits constitutionnellement garantis se dessine quelque chose de beaucoup plus profond, ce à quoi nous attachons une valeur fondamentale, ce que nous estimons devoir être impérativement protégé par notre État de droit, ce qui de manière intangible doit survivre aux tourments et affres du présent, ce par quoi, enfin, nous matérialisons les plus hauts principes de notre République. Certes, la Constitution n’est pas par essence un catalogue de droits, mais ces droits sont le reflet de ce que nous sommes collectivement. Il suffit d’écouter les femmes. » Tel était le conseil prudent, réaliste et sage que prodiguait Simone Veil en 1975. Alors, écoutons les et protégeons les, en constitutionnalisant cette liberté si prompte à être effacée ! La parole

il y a plus d’un an déjà, des femmes du monde entier tournaient leur regard vers la France, plus précisément vers la proposition de loi que ma collègue Mélanie Vogel avait déposée pour constitutionnaliser le droit à l’IVG.

de septembre 2022, la Hongrie décida d’obliger les femmes à écouter les battements de cœur du fœtus avant tout avortement. Ce n’est donc pas un hasard si ce sujet a été porté par une sénatrice représentant les Français établis de France. Tous les ans, nous réclamons davantage d’informations de la part des consulats sur les réglementations locales pour les Françaises de l’étranger et pour les rapatriements de Françaises qui résident dans des pays où elles n’ont pas accès à l’IVG. De nombreuses femmes partout dans le monde s’exposent à tous les dangers – médicaux, légaux, sociétaux… – pour avoir accès à une IVG. Nous pensons à toutes celles qui meurent ou sont grièvement blessées. On peut bien sûr continuer de s’autocongratuler : la France, pays des droits humains, ne serait pas sujette à ce type de régression des droits des femmes. Il suffit pourtant de lire les courriers que beaucoup d’entre nous avons reçus, les nombreuses attaques dont fait l’objet le planning familial, ainsi que celles qui ont lieu partout dans le monde contre le droit à l’avortement. Oui, nous avons besoin de garantir nos droits ! Ce n’est donc pas un hasard si ce sujet est fièrement porté par de jeunes femmes élues au Parlement, nous sommes encore si peu représentées dans les institutions. Je suis heureuse que plusieurs d’entre vous aient écouté les femmes qui les entourent, leurs conjointes, leurs filles, leurs sœurs. Écoutez les, écoutez nous Nous parlons de nos corps, de nos aspirations légitimes. Il est temps aujourd’hui que, en responsabilité, nous votions – que vous votiez – ce projet de loi historique afin de constitutionnaliser la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

Je respecte l’ensemble des points de vue qui ont été exprimés. Je me veux extrêmement modeste, car je n’ai de leçons à donner à personne, à aucun d’entre nous, encore moins au monde entier.

qui ne le seraient pas. À la lecture de la Constitution et de tous les textes constitutionnels, que constate t on ? Le droit de grève : pas garanti. La liberté syndicale : pas garantie. La liberté d’aller et venir : pas garantie. La liberté d’opinion : pas garantie. La liberté de croyance : pas garantie. La liberté d’expression : pas garantie. pas garantie. Le droit de vivre dans un environnement sain – c’est l’article 1 de la Charte de l’environnement – : pas garanti. L’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives : pas garanti

chez le juge constitutionnel – et chez tous les autres juges – un travail d’interprétation qui le conduira à ajouter à ce qui est garanti pour les autres libertés des garanties spécifiques pour celle ci. Cela pourrait mettre en péril l’équilibre entre les droits de l’enfant à naître et la liberté fondamentale de la femme de mettre fin à sa grossesse. C’est la raison pour laquelle je vous demande très sincèrement et simplement que nous fassions ensemble notre travail d’amélioration du texte. On s’en portera bien s’il est adopté après avoir été amélioré.

sera opposable, qu’il donnera lieu à une interprétation, comme vient de le dire le sénateur Bas, du Conseil constitutionnel, dont on ne connaît pas très bien aujourd’hui les tenants et les aboutissants. D’autres pensent au contraire que encore qu’elle renforce la garantie de cette liberté, lui conférant un statut différent des autres libertés fondamentales. Quoi qu’il en soit, la commission des lois du Sénat a considéré qu’il ne fallait pas s’opposer à l’utilisation du terme « garantie ». Elle a donc émis un avis défavorable

et me font dire, et vous font sans doute dire, qu’il a eu mille fois raison de le faire. Monsieur le sénateur Philippe Bas,

Je n’ignore évidemment pas que le terme « garantie » vous déplaît profondément, mais je veux profiter de cet amendement pour tenter de vous réconcilier avec la rédaction du Gouvernement, qui reprend, je l’ai déjà dit et je le répète, quasi intégralement la version votée par le Sénat,

de soupeser avec attention chacun des mots que nous choisissons, cette prudence ne doit pas nous faire céder à une forme de juridisme qui nous détournerait du principal.

Il s’agit d’affirmer dans le texte constitutionnel que la liberté dont il est question est « garantie » à la femme enceinte. Par ces mots, le Gouvernement entend préciser l’intention qui guide la plume du constituant. Il ne faut pas perdre de vue que le texte emporte modification de l’article 34 de la Constitution, exactement comme l’a voulu le Sénat. Or nous savons que l’article 34 de la Constitution est avant tout un article de procédure, consacré à la compétence du législateur. Le terme « garantie » permet de rendre clair le fait que l’objet de cette révision constitutionnelle est non pas simplement d’attribuer une compétence au législateur, qu’il avait déjà au demeurant, mais de guider l’exercice de sa compétence dans le sens du respect de sa liberté. Vous saisissez bien sûr la nuance. Par ailleurs, il est inexact d’affirmer que ce mot est inconnu du texte constitutionnel. On y trouve en fait plusieurs occurrences. La référence la plus évidente se trouve à l’article 61 1 de la Constitution, qui permet à tout citoyen de contester la constitutionnalité d’une loi qui porterait atteinte « aux droits et libertés que la Constitution garantit

Il ne fait en réalité qu’expliciter l’objet et la portée de cette révision : protéger la liberté des femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse. vous rassurer : ce terme ne devrait pas vous inquiéter, car il ne crée en aucune manière un droit absolu, sans limites ou encore opposable.

que la liberté de recourir à l’IVG serait garantie à la femme contre des tentatives législatives de la restreindre drastiquement. Car, oui, le Gouvernement souhaite, en l’inscrivant dans la Constitution, protéger la liberté de recourir à l’IVG. Il souhaite la protéger et non l’étendre. Dans son avis, le Conseil d’État

que, par elle même, l’inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le Gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit,

un instant – « qui sous tend la liberté des médecins et sages femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse ainsi que la liberté d’expression ne crée donc en aucune manière une forme de droit opposable. Pour toutes ces raisons, qui lèvent les incertitudes juridiques, je suis, tout comme la commission d’ailleurs, défavorable à votre amendement.

explication de vote. Je ne suis pas sûre que siffler une sénatrice soit tout à fait à la hauteur du débat.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Alinéa 11 : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Alinéa 13 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » Bref, votre argument, cher collègue,

proposé par Mme Panot de La France insoumise. Cependant, depuis, le Conseil d’État a invalidé cette distinction dans son avis rendu le 7 décembre 2023 et indiqué ne pas faire de différence entre un droit et une liberté : « Au vu de Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne retient pas, en la matière, une acception différente des termes de droit et de liberté, le Conseil d’État considère que la consécration d’un droit à recourir à l’interruption volontaire de grossesse n’aurait pas une portée différente de la proclamation d’une liberté.

peut on considérer qu’il s’agit systématiquement d’une liberté ? Comment doivent le prendre les personnes les plus défavorisées qui y sont poussées par manque de ressources ou par crainte de l’abandon ?

(Drees) conforte, par des études de terrain, la corrélation entre précarité et contrainte d’avorter. Cet amendement spécieux n’a pour but que de masquer votre refus de vous opposer sur le fond à l’esprit général de ce texte. Le terme « garantie » ne fait que renforcer

car le texte perdrait alors tout son sens. L’objet même de ce projet de loi constitutionnelle est bien de protéger les droits des femmes et d’empêcher le législateur futur de les remettre en question.

Or, dès qu’il y a défaillance, le droit recule. La non application de cette loi et les manques en matière de contraception d’urgence expliquent de nombreuses grossesses non désirées et des grossesses précoces, qui peuvent conduire les femmes à devoir avorter. Ce phénomène touche particulièrement mon département, La Réunion, où 12 % des IVG concernent des mineures, soit deux fois plus que dans l’Hexagone.

Il ne prévoit pas non plus une modification de l’équilibre entre les trois principes que vous avez définis et dont nous avons parlé, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté de conscience et la liberté de recourir à l’IVG. En résumé,

le pire n’est pas certain, il est possible. Et nous devons lutter contre le pire dès maintenant, pas au moment où il adviendra. C’est pour cela que nous ne voterons pas cet amendement et que nous souhaitons que cette assemblée vote le texte conforme à celui de l’Assemblée nationale.

la Constitution était uniquement un ensemble de règles juridiques. Or tel n’a jamais été le cas. Juristes et politistes s’accordent sur le fait que c’est également dans la Constitution qu’une société se raconte. Toute constitution, dont la nôtre, retrace aussi l’histoire d’une Nation, parce qu’elle affirme une conception du monde, en énonçant notamment certains droits et certaines valeurs qui se veulent souvent universels. En l’espèce, et cela a déjà été dit, il est évident que la conjoncture politique actuelle, même dans les démocraties occidentales, invite à mettre le droit en position de résistance face à des risques de glissement qui se manifestent partout.

Selon lui, une constitution, c’est l’alliage de deux éléments : d’une part, une « partie efficace », qui assure le bon fonctionnement des institutions

pas d’une querelle de terme. Il s’agit juste de faire en sorte que notre constitution suscite encore plus le respect en protégeant les droits des femmes, de chaque femme, de ce pays.

le terme « garantie » ne crée pas de « droit absolu, sans limites ou encore opposable ». Mais alors pourquoi y êtes vous tant attaché ? Soit, comme l’ont démontré un certain nombre de juristes,

à la jurisprudence. C’est la raison pour laquelle nous préférerions, comme l’a proposé Philippe Bas, que le terme « garantie » ne figure pas

: « En politique, la constance et la cohérence sont vertus. » Avouez, cher collègue, que les vôtres aujourd’hui sont un peu mal en point. c’est que celles et ceux qui, dans cet hémicycle, souhaitent voter pour l’introduction du droit à l’IVG dans la Constitution savent qu’il faut pour cela un vote conforme et qu’ils doivent donc ne pas voter les amendements. Mais celles et ceux qui sont contre l’introduction du droit à l’IVG dans la Constitution,

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

y aurait il eu le 18 juin 1940 ? Y aurait il eu, en 1974, un vote sur l’IVG ? Y aurait il eu, en 1982 ou 1983, un vote sur l’abolition de la peine de mort ? En 1981 ! Et, il y a quelques années, y aurait il eu le vote sur le mariage pour tous ?

la liberté de recourir à l’IVG, qui aujourd’hui n’est protégée par le Conseil constitutionnel qu’en tant que dérivé de la liberté de la femme inscrite à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, il vise à ce qu’il en aille de même de la clause de conscience des médecins, qui découle, elle,

et sur le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, affirme que la liberté de conscience est un « principe

Déjà, en septembre 2018, les sénateurs macronistes, socialistes, communistes et écologistes – la fameuse brochette… – avaient cosigné une proposition de loi de Mme Rossignol

Car, en supprimant l’article L. 2212 8 du code de la santé publique, ils voulaient forcer médecins, gynécologues obstétriciens, sages femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux à ce choix cornélien : violer leurs convictions personnelles, constitutionnellement garanties, ou prendre la porte de leur établissement et de leur profession. Voilà la volonté liberticide clairement exprimée de la gauche. Dans leur marche forcée vers la prétendue émancipation, ils nous passent le carcan ! La menace illibérale est donc bien de ce côté là de l’hémicycle ! Chers collègues socialistes, vous qui scrutez attentivement les discriminations en ce beau monde, n’êtes vous pas capables de voir celles que vous causez par votre idéologie ? Vous devriez vous rebaptiser parti sociétaliste, car vous n’avez rien de social – au contraire, vous piétinez du dépôt de cette proposition de loi de 2018, le Comité consultatif national d’éthique, l’Ordre national des médecins et le Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France se sont opposés à la suppression de la double clause de conscience des professionnels de santé.

Cher Alain Milon, je suis désolé de l’outrance qui est venue au secours de cet amendement et je souhaite reprendre le débat au fond, car le sujet est sérieux.

Or aucune de ces institutions, aucun de ces syndicats de médecins ne tire la sonnette d’alarme ni n’estime que la constitutionnalisation de l’IVG serait une atteinte

médecins. Jamais les femmes qui défendent avec vigueur les droits des femmes ne s’en sont prises à notre clause de conscience. Alors, ne nous en prenons pas à ce progrès pour les droits des femmes

sont les mêmes qui entendent aujourd’hui sacraliser l’interruption de vie dans la loi fondamentale. Cette inscription est manifestement paradoxale et contraire à l’esprit de notre loi suprême. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas ce projet

identique à la version déjà votée au Sénat. Je vais voter ce texte, car j’estime que l’IVG est un droit fondamental pour les femmes. Certains estiment que ce droit n’est pas menacé en France : peut être, nul ne peut le dire aujourd’hui. Nous devons voter la constitutionnalisation de l’IVG pour toutes les femmes qui nous regardent et qui espèrent. Nous devons le faire aussi, car la parole de la France, pays des droits de l’homme, est écoutée, attendue et respectée. Ce vote, c’est aussi un message d’espoir

vous ouvrez la voie à la reconnaissance par le juge constitutionnel, à l’occasion d’une QPC, de l’avortement jusqu’au terme de la grossesse, de l’avortement en raison du sexe ou sur des critères eugénistes. Dire cela est abject ! De même, quelqu’un qui voudrait soutenir la vie à naître pourrait être pénalement sanctionnable face à cette valeur suprême qu’est devenu l’avortement. Tous ces risques en cascade, alors qu’aucun parti ne remet en cause l’IVG, suffisent à fonder mon opposition à ce texte. Une fois celui ci rejeté, nous pourrions valoriser ce qui honore nos principes constitutionnels et civilisationnels, en réfléchissant à une grande politique familiale française incitative par une meilleure protection et un meilleur accueil de la vie.

qui, en 2017, alors ministre de la justice, soulignait l’inutilité d’inscrire dans la Constitution un droit à l’avortement, tout comme François Bayrou et la présidente de l’Assemblée nationale qui, en 2018, affirmait : « Je ne crois pas que la France puisse être suspectée de remettre en cause l’avortement, je ne crois donc pas utile de l’inscrire dans la Constitution.

en indiquant que nous ne pouvions pas faire abstraction de cette difficulté. Pour ma part, constant dans mes convictions, je voterai contre cette inscription d’un droit à l’IVG dans la Constitution. La parole

Notre rôle est de veiller à ce que la rédaction de ce projet de loi constitutionnelle soit la plus intelligible et la plus claire possible, de sorte qu’elle ne donne lieu à aucune interprétation. Nous

parfois mis à mal par la désertification médicale, la diminution du remboursement des actes médicaux, le manque de prévention, d’éducation et de sensibilisation ou encore le manque de moyens des centres de santé sexuelle. Si nous prenons acte du souhait d’une majorité des sénateurs de faire figurer l’IVG dans la Constitution, les membres du groupe Les Républicains voteront chacun selon leur intime conviction. Sans surprise, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera cet article unique et donc le projet de loi.

qui fait sien ce principe fondamental : oui, nous disposons de notre avenir ; oui, nous disposons de la capacité à donner vie, à éduquer, mais celle ci ne peut et ne doit pas être imposée.

Vogel, pour explication de vote. Nous allons faire bientôt un pas immense en France pour la protection des droits et des libertés fondamentales, en énonçant solennellement qu’il n’est pas de société libre, démocratique et égalitaire sans la protection du droit des femmes à disposer de leur vie. Cette immense avancée, nous la devons évidemment aux sénatrices, aux députées, à tous les parlementaires qui se sont battus pour que nous arrivions ce soir à voter en faveur de l’introduction du droit à l’IVG dans la Constitution. Mais nous la devons aussi et sinon surtout à la mobilisation massive de toutes les féministes, de toutes les associations féministes de France, de toutes les femmes, de toutes vos femmes, vos filles et vos nièces,… Arrêtez avec cet argument ! … de toutes les femmes qui sont en tribune ici et qui nous regardent.

Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page de l’histoire du droit des femmes. Ce vote est historique : la France sera le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution Constitution la liberté des femmes à disposer de leur corps. Ce vote, au fond, redit, à ceux qui ne le sauraient pas encore, que les femmes de notre pays sont libres. Ce vote réaffirme à quel point nous sommes tous attachés à cette liberté. Je remercie toutes celles et tous ceux

Merci,